mes chers collègues. Par lettre en date de ce jour, le gouvernement demande de compléter l'ordre du jour du mercredi 14 décembre par l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur acte donner de cette demande, l'ordre du jour appelle l'examen des crédits de la mission cohésion des territoires et article 41, terre du projet de loi de finances pour 2023 et la parole est à monsieur Jean Baptiste, rapporteur spécial de la commission des finances pour sept minutes chers collègues. Madame, madame la présidente, madame la présidente, monsieur le ministre, mes, mes chers collègues, les crédits de la mission cohésion des territoires sont dans le projet de loi de finances pour 2023, 2 17 9 milliards d'euros, l'augmentation des crédits par rapport aux crédits totaux, ouvert en 2022 de 411 millions d'euros, mais cela correspond à une diminution de 1,9 % en euros constants, compte tenu de la prévision d'inflation élevée en 2023 je vous présente les 4 programmes qui porte les crédits destinés aux politiques d'hébergement, d'aide au logement d'urbanisme, de l'habitat, ainsi qu'à la politique de la ville ont constats essentiels sera que ce budget présenté sans que le gouvernement avait présenté des objectifs clairs et tracer une ligne, je le constate sur le programme 177 hébergement parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables, qui porte la politique d'hébergement et d'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, les crédits demandés pour 2023 sur le programme 177 sont de 2,8 milliards d'euros, ce qui correspond en fait à une diminution en euros constants par rapport à 2022 si on prend en compte les crédits ouverts en cours d'année, une fois de plus sur le programme 177 entame l'année avec des crédits qui pourrait bien apparaître comme sous-évalué en cours d'année, et ce d'autant que le gouvernement n'a toujours pas défini d'objectifs clairs pour la politique du logement d'abord, laquelle était une priorité du quinquennat précédent cette navigation à vue est encore plus évidente pour la politique d'hébergement d'urgence car le logement d'abord malgré ses vertus n'a pas permis de réduire le parc d'hébergement d'urgence toujours située à un niveau historiquement élevé, proche de 200000 logements, ce niveau est un plateau dont il semble impossible de redescendre, puisque le gouvernement a renoncé à l'objectif de réduire de 14000 places ce parc en 2023, les raisons sont multiples et il est difficilement envisageable de remettre à la à la rue, les personnes qui ont été hébergées pendant la crise sanitaire, la question des migrants se poser également le dispositif national d'accueil géré par le ministère de l'Intérieur est saturé et engorgent par voie de conséquence, le dispositif d'hébergement du programme 177 le programme 109 aide à l'accès au logement qu'on prend à titre principal les crédits destinés au financement des APL, les crédits demandés pour 2023 sont de 13 4 milliards d'euros et les APL contribue de manière importante à réduire le taux d'effort des des ménages modestes, nous le savons, mais sur le long terme, les prestations sociales couvrent parfois une part de plus en plus réduite des dépenses courantes des ménages et les dépenses de logement augmente, les ménages doivent faire face au poids croissant de l'inflation, malgré les mesures du type bouclier tarifaire, le programme 135 pour sa part, porte des crédits consacrés à des actions diverses liées à la construction et à l'habitat et ces crédits sont de 781 millions d'euros en autorisations d'engagement, soit une hausse de près de 50 % par rapport à 2022 liée au financement de la rénovation énergétique, le secteur de la construction fait face à des tensions sur les prix importante mais aussi aux difficultés toujours élevé à obtenir des permis de construire, tandis que la remontée des taux risque de freiner également la demande, l'autre grand défi est-ce est celui de la rénovation du parc existant, la subvention à l'Agence nationale de l'habitat Pass 170 millions d'euros à plus de 400 millions auxquels s'ajoutent 700 millions provenant des ventes de quota carbone et de 3 milliards sur sur le programme 174 et la mission Écologie pour ma prise rénovent toutefois, il ne suffit pas d'augmenter les crédits pour colmater les brèches des maisons mal isolées, il faut aussi agir sur la structuration de l'offre car il manque un véritable écosystème de la rénovation globale des logements, il faudrait plus d'entreprises capable sur le marché de la rénovation des logements privés, il faut certainement développer mieux les dispositifs qui garantissent une amélioration de la performance énergétique et apporte un accompagnement à des ménages qui n'ont pas la compétence de maîtrise d'ouvrage pour des rénovations globales, or le gouvernement se contente pour l'essentiel d'abonder les crédits de l'aide MaPrimeRénov'de base, certes plus facile à mettre en oeuvre pour publier les chiffres de réalisation impressionnant mais dont l'efficacité n'est pas suffisamment prouvé, s'agissant des logements sociaux, l'objectif de 250000 logements sociaux en 2021 et 22 annoncé par le précédent gouvernement a été oublié et on arrivera peut-être à 190000 sur 2 ans aujourd'hui, les objectifs du gouvernement en matière de logement social, manque de clarté, alors même que le secteur fait face à la hausse importante du taux du Livret A sur lequel ses intérêts d'emprunt centaines d'indexer Action Logement et soumis à une pression hein de pressions importantes particulière d'une part, l'article 16 du projet de loi de finances, le soumis à une contribution de 300 millions pour pour financer les aides à la Pierre, que le Sénat a supprimé d'autre part, et c'est sans doute encore plus important, sa filiale financière Action Logement service a été classé par l'Insee en administration publique risque donc d'être interdite d'emprunt sur plus de 12 mois c'est une décision comptable qui risque d'affecter la participation d'Action Logement aux politiques publiques, dont la mise en oeuvre dépend de sa contribution, à commencer par le nouveau programme de renouvellement urbain, ce programme 135 en toute logique devrait également contribuer au financement du zéro artificialisation nette donc le fameux Anne, ce n'est malheureusement pas le cas indirectement via la dotation cet établissement public foncier sur ce point encore, le gouvernement n'affiche toujours aucune stratégie pour définir un modèle économique Dusan le Fonds friche qui a été très apprécié en 2021 et 22 s'est désormais fondu dans un fonds Vert de la mission Écologie développement et mobilités durables, c'est-à-dire que ni les modalités ni les modalités d'attribution des crédits ne sont connus à ce jour, c'est un flou très regrettable car il entraîne un risque de démobilisation dans un domaine où la vision de long terme est essentiel de manière générale, est essentiel que le gouvernement s'empare réellement de la question du financement et de la fiscalité de l'objectif than afin que les communes, ils voient une opportunité et non une contrainte imposée de manière descendante, j'en arrive, pour finir à la politique de la ville, porté par le programme 147 ces crédits sont de 598 millions d'euros en crédits de paiement en augmentation de 40 millions par rapport à la loi de finances initiale pour 2022 mais quasiment constant en euros constants de ces crédits budgétaires sont principalement consacrée à une grande diversité d'action engagée dans le cadre des contrats de ville mais les résultats de cette politique sont toujours aussi difficiles à percevoir plus de 40 % des adultes de 15 à 64 ans résidant dans les quartiers de la la politique de la ville reste à l'écart du marché de l'emploi, contre moins de 30 % dans les autres quartiers des mêmes unités urbaines pour conclure il faut regretter que le gouvernement cette année encore, repousse le moment où il apportera des financements promis au nouveau programme de renouvellement urbain, qui dépend donc des contributions d'Action Logement et des bailleurs sociaux, alors que les dépenses de l'ANRU commence à devenir importante dépasse dépassant les 500 millions dès 2022, cela n'est pas fait pour nous rassurer, compte tenu des incertitudes pesant sur ces acteurs, le point commun à toutes ces analyses et que ce budget ne présente aucune perspective claire sur le la politique du logement et de l'urbanisme dans les années à venir, et c'est la raison pour laquelle la commission des finances, a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat sur le vote des crédits de la mission cohésion des territoires, elle a en revanche donné un avis favorable à l'adoption de l'Arctique 41 terre qui permet d'éviter un risque d'augmentation de la réduction de loyer de solidarité pour les bailleurs sociaux, je vous remercie. Merci beaucoup, la parole est à monsieur Bernard Delcros, rapporteur spécial de la commission des finances pour sept minutes également. madame la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, il me revient d'évoquer le volet à dominante rurale de la mission cohésion des territoires avec les programmes 112 et 162 qui rassemble notamment les crédits du FNADT le programme 112 voix cette année ses crédits augmenter fortement, de près de 35 %, notamment en raison de crédit rapatrier de l'ancienne mission plan de relance, qui avait été mis en place précédemment, à cela s'ajoutent près de 700 millions d'euros de dépenses fiscales, porté par le programme 112 en faveur de territoire bénéficiant de zonage spécifique, cette version 22023 m'amène à évoquer plus particulièrement 3 sujets. 1er sujet : l'État poursuit sa politique contractuelle avec les territoires, nous soutenons cette stratégie. Les CPER nouvelle génération et les CPER pour les massifs sont désormais signer et opérationnel dans la quasi-totalité des régions, ils bénéficieront pour 2023 de 143 millions d'euros en à eux et près de 56 millions d'euros en CP et de près d'un milliard d'euros sur la période des contrats 2022 2027. Les CRT signé à l'échelle locale et piloté par la haine, c'était entrent dans leur 3ème année de mise en oeuvre, je veux saisir cette occasion pour rappeler que les certes et signé à l'échelle locale doivent permettre aux élus de disposer de visibilité sur les financements de leurs investissements pour la durée des contrats, c'est l'objet même d'une contractualisation pluriannuelle, elle doit s'appliquer dans tous les territoires de France le programme Petites Villes de demain venu compléter fort utilement le programme Coeur de ville se poursuit en 2023. Comme nous le souhaitions, la notion de pour 100, sans critères de nombres d'habitants a été retenu pour l'éligibilité des communes c'était essentiel parce que le statut de pôle de service pour un bassin de vie n'est en aucun cas corrélé à son nombre d'habitants. programme Coeur de ville programme Petites Villes de demain, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de cette logique territoriale de test stratégique que nous approuvons de soutien aux territoires en mettant en place un programme Village d'avenir destinés à l'échelon communal, pourquoi, pourquoi, parce que cela permettrait d'accompagner les territoires jusqu'au plus proche des habitants et d'ouvrir des perspectives aux nombreux maires de petites communes rurales qui se sentent exclus des dispositifs existants, le plan ruralité que prépare la ministre en charge de la ruralité, pour donner une suite à l'agenda rural me semble être la bonne occasion pour mettre en place ce nouveau dispositif et faire aboutir finalement cette stratégie de soutien au territoire 2ème sujet : l'agence nationale de cohésion des territoires bénéficiera en 2023 otite du programme 112 d'une subvention pour charges de service public de 63 millions d'euros, l'agence a aujourd'hui démontré son intérêt même si elle a encore besoin de renforcer sa visibilité à l'échelle territoriale. Elle a bénéficié en 2022 du : hausse de 13 emplois sous plafond c'était nécessaire. Au travers de la haine, c'était le projet de budget pour 2023 maintient les crédits à l'accompagnement des collectivités rurales en matière d'ingénierie. à travers les chefs de projets, des programmes PVD coeurs de villes et territoires d'industrie, les volontaires territoriaux en administration, les chargés de mission fabrique de territoire, les conseillers numérique ou encore les marchés ah bon de commande lancée par l'État, qui présentent un réel intérêt pour le territoire, je rappelle que ces crédits de soutien à l'ingénierie internes et externes, c'était important et nous le demandions, de 10 millions d'euros à la création de la haine, c'était il y a 2 ans, ont été doublés en 2020 21 pour être porté à 20 millions d'euros, comme nous l'avions demandé l'agence pilote également le déploiement de 2500 maisons France services auquel sont consacrés, près de 37 millions d'euros en 2023 et de nouvelles maisons devraient voir le jour dès l'année prochaine, après cette première phase réussi pour les maisons, France, service, nous devons engager une nouvelle étape avec pour objectif une offre de services enrichis l'entrée de nouveaux opérateurs des agents mieux formés et au métier davantage reconnu l'accès à tous les habitants facilité et le financement des maisons pérenniser et revalorisée. Telle est le chantier à mener en 2023 avec le ministre de la transformation de la fonction publique, désormais en charge des maisons rends service enfin j'en reviens aux dépenses fiscales, porté par le programme, sans doute, je l'ai dit, près de 700000 700 millions d'euros, elles sont associées à plusieurs zonage, 7 au total. Ces zonages qui arrivait à échéance fin 2020 ont été utilement prorogé jusqu'à fin 2023, comme nous l'avions souhaité l'année qui vient, sera donc déterminante quant à l'avenir de ces dispositifs parmi eux je veux rappeler ça n'étonnera personne, l'attachement de tous les ruraux au maintien des zones de révélations rural, les fameuses ZRR et au soutien qu'elles apportent à l'économie au secteur médico-social aux collectivités leur maintien est une nécessité pour le secteur rural, je tiens à insister sur ce sujet concernant le programme 162 Interventions territoriales de l'État, il est doté pour 2023 de près de 86 millions d'euros en à E et 62 millions en CP au delà de la reconduction dès 8 actions déjà inscrite en 2022, le projet de budget pour 2023 prévoit une nouvelle action consacrée à la mise en oeuvre du plan de lutte contre les Sargasses aux Antilles, doté de 5,1 millions d'euros, chers collègues, concernant les programmes dont j'ai la charge 112 et 162 je suis assez de personnel, favorable à l'option de leur crédit, mais je rappelle que le vote sur la mission et global est inclus dans le volet qu'a présenté mon collègue Jean-Baptiste Leblanc et sur l'ensemble de la mission, comme il l'a rappelé, la commission des finances a majoritairement et vie émis un avis de Chazey de sagesse, Merci, cher collègue, la parole est à Madame Dominique Estrosi Sassone, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques pour trois minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur spécial le budget pour le logement qui nous est proposé prolonge plus les orientations antérieures qu'il ne fait de choix, c'est un budget de transition qui nous laisse soient inquiets, soit sur notre faim, cet entre-deux est particulièrement sensible sur 3 dossiers clés : le financement du logement social, la rénovation énergétique et la construction neuve, concernant le financement du logement social, l'État a décidé de prolonger la réduction du loyer de solidarité, la RLS d'une année supplémentaire avant toute négociation d'un pacte de confiance avec les bailleurs sociaux ou d'une convention quinquennale avec Action Logement, ainsi, l'article 16 du PLF avait pour but de prélever une nouvelle fois 300 millions d'euros à Action Logement, tandis que l'article 41 terre maintient le rendement budgétaire de la RLS à 1 virgule 3 milliards d'euros, pourtant il n'y avait rien de naturel à cela le Fonds national des aides à la Pierre, le FNAP n'a-t-il pas vocation à être financés par l'État plutôt que par les bailleurs sociaux, la RLS n'a-t-elle pas vocation à disparaître ou pour le moins à décroître face à la hausse des taux d'intérêt des coûts de construction et aux enjeux de rénovation HLM pour un Ministre du logement n'est-ce pas mener une politique à courte vue que de laisser le ministère du Budget prendre de fait le contrôle de 1 % logement demain, Monsieur le Ministre, qui financera la rénovation urbaine ou Action coeur de veille de villes qui sont des programmes vitaux pour les collectivités territoriales, la rénovation énergétique des logements et le 2ème grand sujet, la loi climat et résilience a imposé un calendrier resserré qui est susceptible d'avoir des conséquences majeures sur le logement, car de très nombreuses résidences principales sont classés E, F ou G, un geste attendu et depuis longtemps proposé par le Sénat, a été fait dans le PLFR avec le doublement temporaire du déficit foncier pour les propriétaires de logements énergivores le PLF propose une augmentation importante des crédits de l'Lana mais Monsieur le Ministre donnez-vous pour autant les moyens aux Français de se lancer massivement dans des rénovations globales qui leur permettront de faire des économies précieuses, y compris lorsqu'ils habitent en copropriété, avez-vous entrepris une levée systématique de tous les freins à ces travaux, car c'est toute une filière qui doit se mettre en mouvement, quant au soutien à la construction neuve quelle visibilité allez- vous donner le logement, nous le savons tous est un secteur de temps long et d'investissement qui a besoin d'un cadre stable et tout à l'opposé de niches fiscales prolongé d'une année sur l'autre, ce cadre, je l'appelle de mes voeux pour l'investissement locatif par exemple à travers un statut du bailleur privé je souhaite également que soit réhabilitée l'acte de construire auprès des mères et de nos concitoyens, en sachant lier la capacité financière à agir avec la dynamique de construction de la population sortons enfin de l'absurdité de vouloir construire moins pour loger plus et répondons vraiment aux besoins des Français dans ce contexte, la commission des affaires économiques, a décidé de s'abstenir, elle n'a pas voulu afficher une opposition face à des compromis qui pourrait être constructif, mais elle n'a pas voulu donner non plus l'après-Seconde ça soutenir des qu'elle ne partage pas.

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs spéciaux, mes chers collègues, le gouvernement propose pour 2023 des crédits dédiés à la politique de la ville a d'augmentation de 7,1 soit 39,6 millions d'euros de plus, c'est d'autant plus positif que cette hausse s'inscrit dans un effort quasi constante depuis 2017, c'est d'ailleurs cette constance, ce que je voudrais souligner, de fait, il n'y aura guère de moyens vraiment nouveau, car l'essentiel servira à financer le dispositif, quartiers d'été à hauteur de 30 millions d'euros, qui est déjà en place depuis 3 ans et à une enveloppe supplémentaire de 5 millions d'euros pour des postes d'adultes relais qui sont face et être déjà officiellement ouvert par ailleurs le budget conforte l'ensemble des actions préalablement lancé notamment les 200 cités éducatives pérennisé jusqu'en 2027 et les bataillons de la prévention, ceci étant je ne veux pas minimiser notre satisfaction les quartiers d'été sont confortés et leurs moyens budgétés dès le début d'année, alors que, depuis leur création, à l'issue du confinement en 2020, leur financement n'était assuré qu'en cours d'année, et parfois très tardivement, mettant les collectivités et les associations dans une situation très délicate, ce dispositif était pourtant bé plébiscité par les maires, en raison de son n'aime pas positif en terme de tranquillité publique et d'éducation, je serai plus critique concernant les adultes relais en raison du décalage entre les annonces officielles qui ont porté le nombre des postes sensés être ouverts de 4000 à 6514 au cours du quinquennat précédent et la réalité de 4600 personnes réellement à l'oeuvre sur le terrain, je voudrais Monsieur le Ministre, que vous vous attaquez vraiment aux causes du problème car on sait que la présence au plus proche des habitants est une des clés de la réussite de la politique de la ville, en fait, je voudrais insister ne nouvelle fois sur la situation de l'ONPV pourtant central pour l'évaluation, vous le savez, notre commission a dénoncé le fait qu'il soit devenu une coquille vide, sans personnel sans moyens et sans lien avec la recherche, ou presque, où en êtes-vous de sa relance, Monsieur le Ministre, enfin je veux évoquer la contribution budgétaire l'de l'État au NPNRU, le programme est entré en phase active la rue va donc devoir avoir un rythme de décaissement de l'ordre d'un milliard d'euros par an au cours des 5 prochaines années, or l'État ne tient pas ses engagements, il doit financer un virgule 2 milliards d'euros sur les 12 milliards du programme d'ici 2031 de 2002 7 à 2022 malgré sa promesse d'apporter 200 millions d'euros, 92 millions ont été versés reste donc plus d'1,1 milliard d'euros à payer, soit un rythme de 110 millions par an environ, or une nouvelle fois en 2023, l'État ne versera que 15 millions c'est la crédibilité de l'État qui est en jeu, là aussi, Monsieur le Ministre, nous attendons des engagements en conclusion si je relève positivement la constance du gouvernement dans les politiques menées et les moyens accordés à la politique de la ville, les limites que j'ai indiqué les inquiétudes pour l'avenir, alors que se préparent les futurs contrats de ville ont conduit la majorité de la commission des affaires économiques, a proposé de s'abstenir sur les crédits de la mission cohésion des territoires. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Alain Dufour, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales pour 3 minutes.

bah, présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, le programme 177 des structures d'hébergement qui permet de de lutter seul contre sans-abrisme le l'homme au total des places d'hébergement. Financée constitue l'Open de l'examen de ce programme est absent de 98 % des crédits ne parle d'hébergement a culminé à un niveau inédit de plus de 203000 places en mars 2021, 40000 places de plus qu'en février 2000 y a le printemps 2021, le gouvernement avait fait part de son intention de maintenir de 5000 places ouvertes jusqu'au 31 mars 2022 avant qu'une décrue progressive ne soit amorcée au cours de de cette année pour Antenne 2 le seuil de 186000 E place en 2023, le gouvernement a renoncé néanmoins à son projet de réduction du nombre de places et le programme 177 a été abondé de 40 millions d'euros supplémentaires ce soir va permettre de répondre à l'urgence, alors que la demande de des places est encore très forte, mais nous le savons, la lutte contre le sans-abrisme doit passer d'une réponse construite dans l'urgence, s'appuyant majoritairement sur des places d'hébergement un accès le plus rapide possible logement avec eux donc accompagnement social adapté aux besoins, c'est le sens du plan logement d'abord qui arrive à son terme cette année, ce plan fait l'objet d'un consensus dans le secteur, ces objectifs sont partagées par tout le secteur associatif depuis le le lancement du plan quinquennal à 2017 390000 personnes hébergées aux sans-abri ont accéder au logement social alors une ou à une solution de logement adapté, avec des résultats un MBA continue c'est sorti vers le logement n'ont toutefois pas permis d'enregistrer une baisse de demandes d'hébergement d'urgence, il faut savoir quand même qu'en 10 ans, les crédits alloués au programme ont doublé et ce qu'on ne consacrés à l'hébergement d'urgence ont été multipliés par 4, monsieur le Ministre ou en attendant l'annonce la prochaine séquence du plan logement d'abord dans les délais les problèmes cette mission fait ressortir un problème récurrent, qui n'a jamais été abordé, c'est celui de l'immigration, alors pourquoi je dis ça car sur les 200000 places qui sont, qui ont été attribués bien 15 % sont des nationaux, le reste des personnes sont en situation irrégulière, sans titre ou sans papiers ou en passe d'être expulsés, voilà, situation que je voulais aujourd'hui vous décrire, étant précisé que au regard des moyens financiers qui sont proposés, mais la commission des affaires sociales de sous cette remarque a émis un avis favorable à l'adoption de ces crédits. Oh merci, merci, cher collègue, la parole est à Louis-Jean de Nicolaï, rapporteur pour avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour trois minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, a émis un avis d'abstention à l'adoption des crédits des programmes 112 et 162 compte tenu des faibles évolutions constatées par rapport au budget pour 2022, dans le contexte actuel d'inflation et de fragilisation croissante de l'Agence nationale de la cohésion des territoires 1er point, s'agissant de la société, je relève que l'agence atteint la grande majorité des objectifs qui lui avaient été assignés toutefois, je crains que les financements deviennent ne lui permettent pas de remplir pleinement sa mission de soutien l'IGN sur mesure des communes qui avait justifié sa création dans le cadre de la loi que notre commission avait examiné en 2019, il ne faudrait pas que l'Agence ponctionnent la ligne budgétaire de 20 millions d'euros prévus pour ce soutien à l'ingénierie du fait des contraintes qui s'imposent sur son fonctionne dès lors, il y a 2 solutions : soit il faut attribuer des moyens de fonctionnement à l'agence, à chaque fois qu'une mission nouvelle lui est confié soit il faut mobiliser ses opérateurs partenaires pour qu'ils apportent à l'agence des moyens de fonctionnement, la prochaine révision des conventions pluriannuelles qui qui lie la haine, c'était à des à ses opérateurs partenaires l'Ademe CEREMA en rue, Anna et Caisse des dépôts, doit permettre de remettre sur la table au sujet de la coordination de l'intervention de ces opérateurs 2ème point, la commission estime qu'il est nécessaire de définir une nouvelle ambition pour les politiques à destination des territoires ruraux, la réforme des zones de revitalisation rurale les ZRR est toujours au point mort et des politiques structurantes pour le territoire doivent être amplifié la nouvelle Mini, chargé des collectivités et de la ruralité, a annoncé la préparation d'un acte de de l'agenda rural et c'est une annonce et bienvenue qui doit être conscrits attiser qui pourrait être prolongé par l'initiative législative et réglementaire, notre commission a récemment formulé des propositions sur le commerce en milieu rural, là je logistique urbaine les déserts Monique médicaux et les ouvrages d'art, nous invitons le gouvernement à s'en saisir, je terminerai justement évoquant la question des ouvrages d'art, des collectivités, et plus particulièrement des ponts routiers, la Commission a publié 2 rapports sur le sujet en 2019 avec Hervé Morin, Patrick Chaize et Michel Dagbert, puis en 2022 avec Bruno Belin aussi nous examinerons tout à l'heure des amendements visant à acter un soutien financier de l'État aux collectivités territoriales, à la fois dans le recensement, le diagnostic de ses ponts, mais aussi et surtout pour les accompagner dans la réparation des ouvrages posant des problèmes de sécurité, le programme pont du CEREMA est une première réponse intéressante mais il faut l'amplifier, trop de maires se sentent démunis sur ce sujet, le chantier est colossal : les besoins de financement en matière de travaux de réparation représente 2 à 3 milliards d'euros uniquement pour les ponts du bloc communal, enfin je défendrai un amendement de commission visant à augmenter dans les propositions modestes le soutien de l'État à la reconquête de la qualité de l'eau en Pays de la Loire, je vous en remercie. Merci, cher collègue, dans la suite de notre discussion, je vous rappelle que le temps de parole. Attribuée à chaque groupe pour chaque unité de discussion qu'on prend le temps d'intervention général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de quinze minutes pour intervenir, alors la parole est à monsieur Éric Gold, hein, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen pour cinq minutes chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, le budget de la mission cohésion des territoires frôlera pratiquement les 18 milliards d'euros de crédits en 2023, ça peut sembler conséquents chaque crédit compte puisque cette mission se caractérise par la recherche permanente de la solidarité d'un côté, garantir à tous le droit de vivre dans la dignité, en permettant l'accès à un logement décent et à défaut à un toit et de l'autre, assurer, dans la mesure du possible, l'équité entre les territoires de la République, la crise de structurelle du logement à laquelle vient se superposer une crise énergétique et une inflation qui s'installe dans la durée, nous préoccupe le foncier continuent de se raréfier, alors que nous devons poursuivre la lutte contre l'artificialisation des sols, les objectifs ne sont pas tenus en matière de production de logements sociaux, le parc de logements existants, privés comme comprend environ 5 millions de passoires thermiques quand la sécurité d'approvisionnement énergétique et 2 ans et de moins en moins garanti, malgré les moyens consacrés annuellement à la politique du logement, soit environ 2 % de notre produit intérieur brut, les loyers et les prix d'acquisition des biens immobiliers demeure très élevé dans les villes, les jeunes et les ménages modestes peinent à accéder à la propriété, la part des primo-accédants modestes n'est que de 21 % nous si tout tiendront donc les amendements déposés, qui visent à rétablir à l'APL accession supprimé en 2018, ce type de mesures devrait être privilégié par rapport aux dispositifs fiscaux pour l'investissement locatif bien plus coûteux pour les finances publiques, le développement de la construction ne peut être une réponse partout, alors que nous disposons dans notre pays de bâti inutilisé car fortement dégradée dont on pourrait accompagner l'acquisition grâce à des aides conséquentes et lisible à la rénovation plus de de continuer à favoriser la dispersion de l'habitat, si la montée en puissance de MaPrimeRénov'doit être salué les rénovations globales ne parviennent pas à progresser, encore faut-il Monsieur le Ministre, ce que l'on n'entrave pas la réhabilitation des logements et la redynamisation des centre-ville historique, composée essentiellement de bâtiments énergivores et dégradé qui se vident de leur habitants notamment en secteur sauvegardé, soit plus pour 100 46 % des communes aussi à titre d'illustration, je regrette que la transformation de l'avis conforme des architectes des bâtiments de France, un avis simple pour l'installation de panneaux photovoltaïques n'est finalement pas été retenu au Sénat lors de l'examen du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et, surtout, l'État doit prendre en main la politique d'aménagement du territoire et pour cela permet aux élus locaux de faire vivre leur territoire. La haine c'était n'est pas à notre sens, dotée de moyens en ingénierie territoriale suffisant le sur mesure pour permettre d'accompagner les élus dans la réalisation de leurs projets, les programmes nationaux tels qu'Action coeur de ville ou Petites Villes de demain sont bienvenues pour les collectivités qui ont été retenus pour les autres, en particulier les communes et les communautés de communes rurales, elles ne parviennent tout simplement pas à monter les dossiers pour réaliser des projets et obtenir des crédits de surcroît 6 millions sur les 20 millions d'euros de l'enveloppe dédiée à l'ingénierie territoriale a été puiser pour financer les chefs de projets, de petites villes de demain or face au crédit ouvert dans le cadre du plan de relance, puis maintenant du Fonds Vert le manque d'ingénierie territoriale et surtout d'un guichet unique, comme cela avait été annoncé par le président de la République, les pénalise et ne peut que générer les frustrations l'Agence fêtera ses 3 ans prochainement, nous sommes persuadés que la déconcentration des concentrations de ses interventions doit être accéléré, là où les besoins sont avérés, le recours à des volontaires territoriaux en administration ne peut constituer une réponse satisfaisante, les crédits sont d'ailleurs sous consommer à défaut de disposer d'un guichet unique auprès de la LCD les préfectures étant bien occupé par ailleurs le recrutement de chef de projet, métier qui requiert une certaine expertise serait plus pertinent pour venir soutenir les communes et les communautés de communes rurales dans cette fameuse logique ascendante attendu par les élus, nous présenterons des amendements en ce sens, la transition écologique et énergétique ainsi que la politique d'aménagement du territoire ne pourront être menées à bien sans la pleine participation des collectivités sans une cohésion harmonieuse entre les territoires avec toutes ces remarques, mais au regard des moyens qui seront engagés en 2023, le groupe RDSE votera les crédits de cette mission. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Stéphane Sautarel pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Madame Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, messieurs les rapporteurs, la mission cohésion des territoires comprend plusieurs programmes autour de 2 grands volets : la politique des territoires, sur laquelle je m'arrêterai plus longuement avec des programmes spécifiques qui doivent encore renforcer leur lisibilité pour une plus grande efficacité, une ambition accrue et celle du logement et de l'urbanisme, les programmes 112 et 162 qui concerne la première de ces politiques constitue un des volets de l'action territorial qui figure dans le budget de l'État si les moyens accordés à la haine c'était dont 20 millions d'euros sont consacrés à l'appui des projets portés par les territoires sont stables hors plan de relance, il est bien évident qu'ils ne répondent pas à l'intégralité des besoins de nos territoires, c'est pourquoi il m'apparaît que d'une part, il conviendrait pour renforcer l'ancrage local de la haine, c'était d'expérimenter un appui partenarial renforcé avec les agence technique départementale qui en proximité sont les premières interlocutrice des collectivités et d'autre part de limiter notre corset réglementaire et normatif pour faciliter l'émergence des projets dans des délais raisonnables, il faut en effet sortir du système d'autorisation préalables généralisée pour toute décision que nous connaissons,

coalisées une somme de documents qui sont opposables en droit et tout ça effectivement et générateur de temps de délai qui ne sont plus toujours compris cela oblige à avoir une ingénierie technico-juridiques, administratives qui amplifie les fractures territoriales en voir un incluant certaines collectivités qui n'ont pas les moyens, nous devons absolument redonner confiance dans nos procédures, le réseau France, service, quant à lui est proposé en stabilité de crédits à hauteur de 36,3 millions d'euros, nous arrivons en effet en vitesse de croisière du déploiement de ces maisons qui bénéficient d'un forfait d'accompagnement financier à hauteur de 30000 euros je veux saluer le travail de notre rapporteure spéciale : Bernard Delcros très investi sur cette action qui a conduit une mission de contrôle éclairante, confirmant la pertinence du dispositif mais aussi certaines limites et quelques pistes d'amélioration, notamment quant au renforcement de leurs Liens avec les communes du territoire, à ce titre, je soutiens la démarche visant à accroître le forfait à louer pour tendre vers une participation à 50 50 l'objectif serait de parvenir à une participation de l'État a en effet et de ses opérateurs de 50000 euros au titre de ses missions de service public national assurées par les communes et les EPCI qui ne nous est pas possible durablement de mobiliser au-delà de la moitié du coût, qui s'établit à 100 ou 110000 euros, passé de 30 à 35000 euros de forfait contributif en 2023 serait déjà une première étape. Enfin, la question sensible des zonages, et en particulier des ZRR doit être rapidement traitées pour donner lisibilité et garantie si on peut se féliciter d'une prorogation du système actuel jusqu'au 31 décembre 2023, comme ça a été rappelé, il est clair qu'il faudra très vite harmoniser le zonage adapter les mesures sur la base de l'évaluation réalisée et sans doute introduire des mesures nouvelles de valorisation renforcé des aménité rural qui serait plus positive encore concernant le volet logement et urbanisme qui concerne 17 9 milliards d'euros en plus de la dépense fiscale de 15 9 milliards et des ressources affectées je me contenterai d'une seule observation qui constitue aujourd'hui l'inquiétude majeure sur tous nos territoires ruraux, il s'agit bien sûr de la mise en place du qui doit être assouplie territorialisée et différencier la mission de contrôle transversales et transpartisane sous l'égide de notre collègue Jean-Baptiste Leblanc qui rendra je crois, c'est ses conclusions et des propositions sous une dizaine de jours devraient être éclairante de ce point de vue là et j'espère qu'elle sera entendue, il s'agit à la fois de rendre au maire la capacité à maîtriser l'aménagement de leur territoire aux territoires ruraux à ne pas être victime de la double peine, à savoir avoir peut consommer d'espace dans le passé et donc avoir encore moins de besoins d'équipement d'une part et d'autre part, devoir être les plus gros contributeurs à la non-artificialisation des sols, ils doivent garder une capacité à agir dans nos territoires, mes chers collègues, ne manqueront malheureusement probablement d'agriculteurs avant de manquer de terrains agricoles, il faut donc que l'espace qui est notre richesse soit maîtrisé par les acteurs locaux je interviendrait dans le débat sur cette question qui me semble essentielle et sur laquelle nous devons donner des gages à nos territoires, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jacques Fernique, pour le groupe écologiste solidarité territoire pour cinq minutes. merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de commission, messieurs les rapporteurs, chers collègues, cette mission budgétaire rassemble des dispositifs relevant de 3 commissions permanentes de notre assemblée, elle traite en partie du logement, de l'hébergement d'urgence, la politique de la ville, des outils de contractualisation entre l'État et les collectivités de l'action de la haine, c'était en appui aux projets territoriaux et d'une série d'interventions territoriale ciblé entre autres algues vertes en Bretagne chlordécone en Martinique, Guadeloupe, une mission assez disparates, mais dont les composants différents nécessite en commun un renforcement des dispositifs de soutien pour contrer les basculement dans la précarité et lever les obstacles, aggravé par les crises au dynamique de nos territoires en transition, disons d'emblée que pour ce qui est de ce renforcement, le compte n'y est pas tout à fait puisque, à périmètre constant, en intégrant l'inflation, les crédits de cette mission devrait diminuer en volume de près de 2 très sommairement dans le temps imparti, voici les principales appréciation préoccupations et propositions de mon groupe, d'abord nous ne discerne ont pas vraiment dans les 3 programmes dédiés au logement, une vision politique et des orientations nouvelles conséquente, répondant à l'ampleur du mal logement régulant de façon volontariste les prix tendu loyer que du foncier procurant aux bailleurs sociaux, les marges de manoeuvre à la hauteur des besoins criants permettant aux primo-accident aux primo-accédants aux étudiants et aux jeunes couples d'accéder au logement dans les coeurs de nos métropoles et les zones touristiques colonisé par Les Herbiers Bill et résidences secondaires, les locations saisonnières et de trop nombreux de logements vacants, face à l'absence de réelle volonté d'y répondre par des crédits à la hauteur, mon groupe votera bien sûr les amendements visant à améliorer les APL et dès l'accession à la prison, propriété des ménages modestes, réduire les logements inadaptés aux personnes dépendantes hébergées les les femmes victimes de violences, pour ce qui est de l'hébergement d'urgence, la forte tension a obligé le gouvernement à annuler la réduction prévue de 14000 places face à l'ampleur du nombre de personnes de familles d'enfants à la rue, survivant dans des conditions indignes dans nos grandes villes, notamment à Strasbourg, l'État ne peut laisser sans appui réel nos collectivités en première ligne face à ces drames humains sur lesquels les engagements au plus haut niveau n'ont pas été tenues les collectivités souhaite travailler sur ces hébergements d'urgence avec un État réceptif à leurs propositions, avec un État facilitateur, on y arrivera mieux sur le front du logement encore la vraie nouveauté, c'est le renforcement des moyens de l'Lana pour la rénovation thermique, la dernière note de France Stratégie convaincra sans doute ce qui n'avait pas pris toute la mesure du gouffre énergétique qui est notre parc résidentiel MaPrimeRénov'prend certes son ampleur, mais son bilan énergétique avéré, hé bien plus réduit, il représente pour l'instant 0 45 % d'économie sur la consommation totale du parc résidentiel, nous sommes encore très loin de rénovation globale mise en oeuvre de manière massifier le groupe écologiste proposera à notre Sénat d'enquêter et de proposer de façon approfondie pour que ces politiques publiques trouve les voix de l'efficacité sur le front des quartiers de la politique de la ville, la persistance d'une pauvreté et d'un chômage nettement plus important oblige à amplifier nos actions publiques le nouveau programme national de renouvellement urbain est entré en phase active si les bailleurs sociaux et Action logement sont au rendez-vous, l'État n'a pas pour sa part tenu ses engagements, soit un rythme de 110 millions par an avec 15 millions pour 2023, ça vient d'être appelé, on en est loin avec un observatoire de la politique de la ville en panne et indigents, on est loin encore d'avoir l'outil d'évaluation qu'il faudrait, au moment où les perspectives financières des collectivités s'assombrissent lourdement ou leur capacité à mener leurs indispensable investissements d'avenir et fragilisé les programmes et dispositifs d'accompagnement à leur profit apparaissent d'autant plus essentiel dans ce contexte tendu, l'Agence nationale de la cohésion des territoires ne peut se borner à une stabilité de ses moyens, au regard de ses missions, notamment pour le déploiement de nombreux programmes nationaux, l'accompagnement en ingénierie des élus pour les aider à concrétiser leurs propres projets, le budget de la une, c'était est manifestement insuffisant, enfin mon groupe et de ce nombre ici qui pensent que l'État doit renforcer sa part de prise en charge des Maisons France service, celles-ci sont des palliatifs utile au recul des services publics dans les territoires de la République, je proposerai d'ailleurs un amendement d'autant les maisons France, service d'une compétence et de moyens pour l'accompagnement et le conseil en mobilité avec l'avènement des ZFE et la décarbonation accélérer les déplacements voilà un service d'intérêt public qui s'impose, puisqu'il me faut conclure, vous aurez compris que le vote de mon groupe, sur les crédits de cette mission sera complètement conditionné au sort qui sera fait aux nombreux amendements nécessaires pour que soient contrer les basculement dans la précarité et lever les obstacles au dynamique de nos territoires en transition. Merci, cher collègue, oui c'est très bien. La parole est à madame Nadège avis pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants pour six minutes. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des finances, mesdames et messieurs les rapporteurs, monsieur le Ministre, mes chers collègues, doté de 60 milliards d'euros dans ce projet de loi de finances pour 2023, les ministères de la transition écologique de la cohésion des territoires de la transition énergétique voient leur budget atteindre un niveau inédit des moyens d'ampleur face à des défis, nous le savons colossaux, la mission qui nous occupe ce matin entend soutenir la cohésion des territoires en accompagnant les collectivités territoriales dont les ressources sont confortés et en maintenant notre mobilisation en faveur des territoires et des personnes les plus fragiles, les crédits qui sont dédiés sont en hausse de 3 7 % en autorisations d'engagement par rapport à 2000 22 et de 3 9 % en crédits de paiement, je veux revenir tout d'abord sur ce affecté à l'hébergement et au logement, à savoir les programmes sont neufs, 135 et 177 dotés à eux seuls de près de 17 milliards d'euros, il est à noter la progression sensible des moyens alloués à l'Agence nationale de l'habitat qui ont plus que doublé, afin de couvrir la création de 25 postes supplémentaires d'accompagner le déploiement du réseau France rénove et de préparer l'adaptation des logements au vieillissement de la population, avec le déploiement de ma prime adapte de même le budget consacré aux aides personnalisées au logement augmente quant à lui, de près de 300 millions d'euros pour accompagner les décisions que nous avons prises cet été avec la revalorisation des APL, de l'ordre de 3 5 pour lutter contre l'inflation, il se situe à 13,3 milliards d'euros, le programme 177 qui s'élève à 2 8 milliards d'euros et destinés à l'accès au logement pour les personnes sans abri ou mal logées, les capacités d'accueil du parc d'hébergement généralisé, financé par l'État seront renforcés pour atteindre 197000 places d'hébergement l'année prochaine grâce à une enveloppe supplémentaire de 40 millions d'euros, il est aussi prévu le financement de la revalorisation des métiers du secteur accueille hébergement insertion en matière de politique de la ville à travers le programme 147 l'engagement financier du gouvernement se poursuit, là encore, avec une hausse de 7 % des crédits, celle-ci est supérieure à l'inflation anticipée était en augmentation constante depuis 5 ans, les objectifs poursuivent le financement du dispositif Quartiers d'été qui rentre contre un grand succès dans nos campagnes, accompagner la montée en puissance de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi financés des postes d'adultes relais supplémentaires qui permettront à des personnes sans emploi ou bénéficiant d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi d'assurer des missions de médiation sociale et culturelle de proximité, assurer la continuité de plusieurs politique initiée il y a quelques années, et je pense tout particulièrement aux 200 cités éducatives qui sont pérennisées jusqu'en 2027 cela donnera de la visibilité à ces nouveaux cadres locaux de coordination visant à mieux accompagner les jeunes dans leur parcours éducatif de leur naissance jusqu'à leur insertion professionnelle, le programme 112 a quant à lui, fait l'objet pour objet l'impulsion à la coordination de la politique d'aménagement des territoires pour assurer l'égal accès des citoyens à un socle de services fondamentaux je ferais ici référence à 5 actions principales, l'accompagnement des Maisons France service il en existe désormais une trentaine labellisés dans le Finistère et plus d'une 2000 plus de 2000 sur le territoire national, la déclinaison de l'agenda rural à travers notamment Petites Villes de demain, le programme territoires d'industrie, les contrats de plan État-Région ou encore le plan Action coeur de ville dont le second volet vient d'être annoncé le dispositif gouvernemental restera le même, avec un axe environnemental fort et une enveloppe de 5 milliards d'euros sur 4 ans au lieu de 6 de son côté la c'était voit sa subvention pour charges de service public, stabilisé à travers le programme 162, il s'agit de mettre à disposition des acteurs locaux de l'État une enveloppe budgétaire unique fond J. fongibilité en provenance des programmes multiple, plusieurs sont là aussi consacré à Adré bourreaux problématiques environnementales territoriale je citerai la continuité du financement de l'action oh et agriculture en Bretagne, qui vise à réduire le développement des algues vertes ou encore la création d'une nouvelle action afin de lutter contre la prolifération des algues Sargasses aux Antilles 14 communes sont concernées en Guadeloupe et 9 en Martinique, globalement, il s'agit donc de constater une continuité bienvenue des politiques publiques en la matière, celles mises en place depuis 2017 avec une nouvelle fois une dimension environnementale prépondérante notre groupe se prononcera en faveur de ces crédits, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Denis Bouan One pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour cinq minutes. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre. Monsieur le président de la commission des finances, messieurs les rapporteurs, chers collègues, dans son discours de politique générale, madame la première ministre de rappeler que la pub pour la plupart des Français, le logement et la première dépassent malheureusement malgré cette réalité, les politiques du logement n'ont pas fait partie des grandes priorités de la précédente législature, 4 milliards d'euros qui sont prélevés chaque année sur les autres causes OPH à travers la RLS en ensemble la plus criante illustration les bailleurs sociaux alerter sur les conséquences de telles dispositions, une clause de revoyure avaient été décidées, j'entends ceux qui disent que, malgré les secousses de la Sécu, la situation financière des organismes HLM est aujourd'hui stabilisée, j'entends parfois les mêmes discours au sujet des finances des collectivités locales, alors oui, les bailleurs sociaux comme les collectivités sont des choses qui en est responsable, mais à quel prix la construction de logements sociaux, monsieur le ministre a diminué de 36 % en quelques années ce constat dans 12 inciter à sortir cette approche comptable, la simple stabilisation financière nationale qu'on ne peut pas être un objectif suffisant à l'heure où plus de 2 millions de Français sont dans l'attente d'un logement social d'urgence de l'inflation ne doit pas 12 empêcher d'agir durablement pour le pouvoir d'achat des Français à part à travers des politiques structurantes. Le logement pourrait être la première de ces politiques et le logement social, le 1er nouveaux leviers 7 personnes sur 10, il faut le rappeler sans doute éligibles à un logement social y habiter un permis en moyenne une économie de 227 euros par mois à l'heure où le marché de l'immobilier accentue les inégalités mesurons la portée de ces chiffres, nous avons entendu l'annonce à madame la première ministre d'un pacte de confiance avec les acteurs du logement social. Dans le cadre de la remise en place de la FLS serait un bon 1er pas pour dessiner les contours de cette confiance, le fait de reconnaître le logement social comme une politique de première nécessité de vis-à-vis de la nation, soutenant l'ensemble des investissements des organismes HLM à une TVA réduite à un taux de 5 virgule cinq seraient également un très bon signal aussi, je regrette que les amendements que nous avons déposé en ce ça ne sont pas n'ont pas d'été retenu par le ce PLF. Par ailleurs, la flambée du prix de l'énergie n'exige des réponses urgentes et promis l'application sans faille du bouclier tarifaire, elle met également en lumière la la nécessité d'accélérer la rénovation énergétique de logements en priorisant ménages précaire par la mise en place d'un prêt à taux zéro il faut favoriser les travaux plus ambitieux pour qu'fait en perçoivent les signes concrets d'une sans transition énergétique trop inefficace, trop inégalitaire, nous y reviendrons bien sûr dans le débat s'agissant du nouveau du nouveau plan logement d'abord quelles seront les orientations et surtout quels seront les moyens pour apprécier l'accompagnement social encore trop insuffisants pour les plus précaires, à contrario, certaines dans nos amendements ont été retenus, certaines mesures vont dans le bon sens Monsieur le Ministre, je pense à ma prive adapte qui favorisera la natation, dire aux chômeurs, vieillissement de la population et si l'âge, il s'agit là d'un véritable défi pour notre société et nous devons non avait les moyens de le relever, nous sommes donc heureux que cet amendement que nous avons proposé pour en corriger la cohabitation intergénérationnelle et soit retenue, nous sommes également satisfaits de la tempe sont de l'adoption de l'entraînement demain concernant le prolongement du du prêt à taux zéro jusqu'en 2026 c'est un sujet important qu'à l'obtention de crédits immobiliers, de plus en plus contrainte pour les ménages modestes dans la même optique, nous voterons l'amendement qui est porté par reporteur concernant l'APL accession c'est une aide qui est un véritable effet déclencheur pour donnant peu ménage malgré quelques avancées positives, ce budget logement ne démarre se démarque par des politiques menées lors du précédent quinquennat si cela peut s'expliquer, tenu du calendrier nous espérons vivement que le prochaine sera celui de la rupture, de nombreux signaux d'alerte sont aujourd'hui au rouge à ce qui concerne le logement des Français le parcours résidentiel telle qu'il est coincé : quoi, les policiers, la part des ménages propriétaires de leur résidence principale ne progresse plus, la tension entre l'offre et la demande ne cesse de se renforcer le nombre de résidences secondaires et de logements occasionnels augmente plus vite que l'ensemble du parc, en fait la disponibilité du foncier, son prix, qui ont de plus en plus qu'entraîne, y compris dans les territoires ruraux, monsieur le Ministre, face à ce constat, Ronan des sénateurs socialistes, d'autres collègues, le président pas du crâne, nous a rappelé à faire du logement la grave de code national de ce quinquennat nous ne pouvons pas nous satisfaire des dispositions qui sont prises à leur projet de loi de finances 2023, mais nous espérons toujours que cet appel sur et au logement sera demain la grande cause nationale du prochain projet de loi des finances. Merci, sa collègue, la parole est à Madame Marie-Noëlle Lienemann pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste pour cinq minutes. Monsieur le Ministre, madame la présidente, mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, la crise du logement non seulement perdure mais s'amplifie le le logement coûte trop cher, plombe de plus en plus le pouvoir d'achat de nos concitoyens, la construction de logements est particulièrement de logements sociaux ou abordables s'effondre, les logements indignes ne se résorbe pas et même avec le vieillissement du parc, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus dangereux, la résorption des passoires thermiques n'a pas trouvé un rythme de croisière permettant d'atteinte des objectifs de la loi climat-énergie d'une certaine façon, Monsieur le Ministre, vous le reconnaissiez il y a quelques jours, on indiquant, on doit tous se mobiliser pour que le logement ne devienne pas la bombe sociale de demain. Ce budget, répond-il à cette injonction, la réponse était hélas non aucun réel progrès n'y était, il n'y être inscrit pour enrayer cette crise est pire, certains reculs ils sont consacrés d'abord, ce budget ne propose aucune décision qui répare des graves erreurs du précédent quinquennat qu'il s'agisse de l'APL du prélèvement sur les bailleurs HLM avec la MLS le niveau de la TVA pour le logement social, rien pour réguler les dérives de prix, en particulier ceux du foncier qu'il serait grand temps d'encadrer pour stopper cette spirale haussière qui renchérit indument la production de logements accentue la ségrégation sociale et spatiale, il serait pourtant urgent de s'attaquer à la rente foncière. Ce budget ne répond pas non plus et l'urgence sociale et ne prend pas en compte l'impact redoutable de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie, votre gouvernement n'a pas retenu la proposition de gel des loyers que défend notre groupe et a fixé à 3 5 la hausse de l'IRL, soit un niveau supérieur à la hausse moyenne des salaires cette année, de fait, cette décision va pénaliser le pouvoir d'achat d'un grand nombre de foyers les APL ne devraient pas augmenter ne devrait ce qui ne compensent pas la hausse effective de la quittance qui comprend non seulement les loyers, mais aussi les charges locatives, en particulier le chauffage, or ces dernières augmentent très fortement et le bouclier énergétique ne pour ne ne couvre pas l'entièreté de séance de plus de nombreux locataires HLM n'en bénéficient toujours pas, nous regrettons que le forfait charge des APL qui n'avait pas été revalorisée depuis 12 ans ne soit pas fortement augmenté cette année où tout pourtant le justifie les deux euros de juillet ne suffisent évidemment pas, vous auriez pu à cet effet, mobiliser les un virgule 5 millions d'euros économisés par l'État sur le dos des populations modestes avec la mise en place de la côte pour été des APL, sans en revaloriser le niveau refus de taxer les surprofits mais ponction sur les APL et les bailleurs sociaux oui, Monsieur le Ministre, c'est le trou d'une bombe sociale, la hausse du taux du Livret A s'ajoute au maintien de la FLS, dont nous demandons l'abrogation obérant de façon inquiétante les capacités des organismes HLM de construire, rénover, entretenir leur parc ce budget consacrent le total désengagement de l'État dans l'aide à la Pierre pour le logement social qui, pourtant, on a fortement besoin. il en a besoin pour produire plus pour des loyers moins chers et mieux adaptés aux ressources des familles, la Fnac n'est plus, abondé par l'État depuis plusieurs années, mais seulement par les bailleurs sociaux et Action logement si cette année il est maintenu au même niveau que précédemment, ce qui est déjà très insuffisant et ne suit pas l'importante hausse des coûts des travaux, c'est au prix d'un prélèvement de 300 millions sur Action Logement : le Sénat a bien voté un amendement contestant ce prélèvement mais en même temps très clairement signifié qu'il devait être compensée par l'État et qu'il ne saurait y avoir du coup une baisse de la dotation du FNAP le maintien de la dotation du FNAP doit être garantie, c'est pour notre groupe, une priorité absolue et je le crois, pour notre Sénat car le FNAP est le seul outil qui assure vraiment l'égalité d'accès et de subventions pour tous les organismes HLM, quelle que soit leur statut, l'accession sociale à la propriété semble avoir disparu des radars du gouvernement, c'est pourtant tout à la fois une aspiration de nos concitoyens comme un atout pour le parcours résidentiel et dans bien des cas pour la mixité sociale, l'absence d'engagement sur le PTZ au delà de 2023, comprendre ce qu'est le lancement de nouveaux projets, ce n'est pas acceptable et d'ailleurs, j'espère que vous accepterez le l'amendement du Sénat je termine enfin pour dire que la hausse des taux, la restriction de l'accès au crédit, qui pénalise les catégories populaires et moyennes nécessite une prime d'accession sociale pour y remédier, pour l'heure, rien n'est prévu alors dans ces conditions, mes chers collègues, monsieur, madame la présidente, et Monsieur le Ministre, le groupe CRCE ne votera pas ce budget. Merci, la parole est à madame la présidente, Valérie Létard, pour le groupe Union centriste pour huit minutes. madame la présidente, monsieur le ministre, Messieurs, madame, les rapporteurs, mes chers collègues, au-delà du seul exercice comptable et budgétaire, la mission dont nous discutons aujourd'hui, mais c'est aussi valable, plus largement, pour le PLF doit nous amener à réfléchir au modèle de société que nous souhaitons soutenir pour les générations futures et pour notre pays, cette discussion intervient dans un contexte que nous savons perturbés au lendemain d'une crise sanitaire, nos concitoyens doivent désormais faire face à des difficultés liées à l'inflation à la crise énergétique et aux nombreuses incertitudes qui en découlent, ah ces crises vient s'ajouter celle du logement, nous le savons, nous devons relever de nombreux défis, rendre plus sobre nos logements pour atteindre la neutralité carbone continue de construire pour soulager les zones tendues et faire face à la demande en tout territoire et favoriser le parcours résidentiel, source d'épanouissement familial et personnel de nos concitoyens, c'est pourquoi nous entendons rappeler aujourd'hui, au sein de cet hémicycle que le logement, monsieur le ministre, hé bien de première nécessité et non pas une variable d'ajustement des politiques publiques de l'État, à ce titre, nous soutenons les mesures prises dans le secteur de l'hébergement des personnes vulnérables, nous saluons la revalorisation des métiers du secteur accueille hébergement insertion qui représentera 148 millions d'euros de plus en 2023 ainsi que les nouveaux développements en matière de logement d'abord destiné aux plus fragiles à hauteur de plus de 44 millions d'euros, notre pays doit rester fidèle au principe d'accueil inconditionnel, le gouvernement a d'ailleurs accepté d'amender le budget initial de 40 millions pour maintenir les 195000 places d'hébergement Renault 100 ans baisser ainsi le nombre, ce qui veut quand même dire, Monsieur le Ministre, que tout en assurant effectivement ce principe inconditionnel, il faut que l'État mette les moyens et créer les conditions pour qu'il ne soit pas dévoyé et qu'il soit maîtrisé. Ce volume de places qui est augmenté pendant la crise Covid doit être maintenu, il constitue donc désormais un plateau qu'on ne peut restreindre, nous resterons vigilants sur ce point, sur le plan budgétaire des efforts importants sont également réalisés pour la rénovation énergétique des bâtiments et du logement, l'Anaes voit son budget s'accroître de 900 millions d'euros via le programme 174 et 219 millions grâce à l'affectation de recettes de quota carbone dans un contexte où la France se fait rappeler à l'ordre pour son retard en matière de rénovation énergétique des logements, l'Anaes doit renforcer son intervention, rappelons qu'entre 2000 19 et 2021 toutes aides confondues le décaissement du réseau, les décaissements du réseau ont été multipliés par 3 le nombre de logements aidés par 5 concernant MaPrimeRénov', le compte n'y est pas totalement malgré les moyens conséquents, elle a été attribué à 644000 logements 2021 pour un un montant moyen de 3200 euros MaPrimeRenov c'est sérénité a permis même cette année, la rénovation de plus de 41000 logements dont plus de 23 ans 23000 ont bénéficié d'une bonification pour sortie de passoires thermiques MaPrimeRénov'co-prod fait son chemin, avec en 2021 12000 logements concernés

il y a un dernier point sur lequel vous voulez peut être porter votre attention, c'est que si, effectivement, côté MaPrimeRénov', on voit bien que les efforts sont conséquents, il manque malgré tout dans ce dispositif une réflexion véritable pour avoir les mêmes ambitions de massification, qu'il s'agit du crédit d'impôt qui n'est plus là pour les classes moyennes qui sont aujourd'hui en difficulté par rapport à un effort significatif d'accompagnement de la massification de la rénovation des logements et vous dire aussi que sur les enveloppes délégués au préfet de région, il y a des régions, ces enveloppes sont insuffisantes, puisque dans la mienne, il manque 40 millions et nous sommes obligés de rattraper rattraper, année après année, des retards d'instruction de dossiers, il nous faut intensifier aussi donc c'est politiques de sobriété énergétique, les objectifs atteints de son de son aussi confronté à de nombreuses injonctions contradictoires qui sont posées aux acteurs du logement, de l'interdiction progressive de louer des passoires thermiques voté dans la loi climat au 0 artificialisation nette. Et j'associe à ses réflexions bien sûr mon collègue Jean-Baptiste Leblanc en tant que rapporteur. Et sa déclinaison dans nos territoires, la transition énergétique dans notre pays devient trop souvent synonyme d'une vision décliniste du logement à la lecture de ce budget, il nous paraît il nous faudrait construire moins pour loger plus, comme le rappelle notre rapporteur Dominique Estrosi, l'équation est manifestement insolvable, le secteur de la construction de logements neufs étant en grande souffrance, or on ne peut prétendre pouvoir vouloir protéger les générations futures, si on ne le l'air on ne leur laisse pas de place pour se construire leur foyer, il ne s'agit pas là de faire le procès de la transition écologique, bien au contraire, elle est indispensable, il y a le des Erich aux ménage dans la maîtrise de leurs charges et continuerait bien sûr à défendre la nécessité d'agir en ce sujet mais il y a aussi l'objectif poursuivi et sa mise en oeuvre et il y a évidemment la nécessité de marcher sur 2 jambes, la jambe de la rénovation, la jambe de la construction, la mission de contrôle que j'ai l'honneur de présider sur le sujet de la zéro du zéro artificialisation nette avec notre rapporteur Jean-Baptiste Leblanc sera force de proposition aussi sur les ambitions nécessaire à corriger pour faire en sorte que Lausanne et l'acte de construire reste évidemment hé bien nous le voyons ce conflit entre des objectifs de politique publique majeur est aujourd'hui manifeste et les choix politiques opéré là où ils auraient dû et pu s'inscrire dans une logique de développement durable semble avoir omis l'aspect économique et social au profit du seul aspect environnemental, là où ils doivent raisonner ensemble. Au travers de l'examen, on constate cette année une augmentation du financement des APL à hauteur de 292 millions d'euros, il s'agit ici de la traduction des décisions votées cet été dans le projet de loi, pouvoir d'achat qui prévoit d'accroître de 3 5 % les paramètres de calcul des APL. En raison de l'inflation, nous pourrions nous en féliciter, s'il ne s'agit-il, c'est là que d'une mesure de réactions qui nous rappelle avant tout le contexte dans lequel il s'inscrit une crise du logement, cette dernière n'épargne pas le nombre de, le, le monde du logement social aux difficultés déjà malheureusement bien connu, les bailleurs sociaux fragilisés depuis 2018 par la RLS voient leurs difficultés se renforcer normalement en ce qui concerne le manque d'autofinancement, il ne dispose plus des mêmes moyens pour financer les nouveaux programmes de construction la rénovation thermique des logements et donc des risques et leurs locataires multiplient les alertes sur la hausse des coûts de production des taux d'intérêt et l'impératif toujours plus prégnant de rénovation et de construction, nous devons être davantage attentif face à ces signaux et même offensif, Monsieur le Ministre, l'État doit être offensif les doigts, l'État doit reprendre toute sa place. Et financer les politiques du logement plutôt que d'aller chercher les moyens chez les acteurs, qui sont des partenaires, mais qui ne doivent pas être des financeurs. Je alors dans un contexte particulier ou comme je viens de le dire, le secteur du logement vous manque de visibilité, il convient de souligner en plus la pression exercée par le gouvernement sur Action Logement. Action Logement. Mes collègues l'ont tous déjà rappelé mais ce point, il est particulièrement important, c'est pas à vous que je vais la prendre Monsieur le Ministre, vous le savez pertinemment, d'abord il y a 2 2 millions de foyers qui sont en attente de logements sociaux aujourd'hui, donc quand on nous explique qu'il ne faut plus construire, qu'on est en train de décliner sur les demandes bah on peut décliner un moment avant d'avoir de 2 millions de solutions pour les 2, 2 millions de familles qui attendent toujours d'avoir un logement, alors on peut rénover, on peut dire qu'il y a des logements vacants, mais où sont-ils vacants à l'endroit où on en a besoin, je ne suis pas sûr et les décohabitation il y a des territoires dans lesquels ce ne sera pas possible alors, mes chers collègues, Action Logement a besoin, comme nous l'avons fait dans le cadre de l'amendement, qui est passé à l'article 16 Action Logement a besoin bien évidemment d'être soutenu pour être au rendez-vous de la décarbonation, mais enfin Monsieur le Ministre, permettez-moi de vous dire que, il faut sans attendre le PLF de l'année prochaine, envisager un vrai plan de décarbonation, une vraie, un vrai engagement de l'État comme acteur et financeurs du même si son collègue à la hauteur des besoins de ce pays et des 30 % que représentent le monde du logement dans cette politique de décarbonation. Merci, hein, c'était huit minutes ce n'était pas la parole est à monsieur François Bonhomme pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre, ces programmes touche à une question essentielle des moyens à la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de cohésion du territoire, il faut dire préalablement que l'éclatement des crédits qui concourent à cet objectif ne facilite pas une analyse globale des moyens de cette politique, pas plus d'ailleurs que une analyse d'une éventuelle stratégie il faut dire aussi que le fléchage des crédits, je pense à une partie de ceux du plan de relance du ministère de l'Économie complique l'analyse par manque de lisibilité concernant le programme 112 impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire, on pourrait saluer hausse mais celle-ci n'est que de façade, si l'on considère les crédits pour 2000 22 et ceux prévu dans la mission du plan de relance qui ont été transférés en gestion à ce programme 112 c'est bien une baisse qu'on constate, attends un acte d'engagement qu'en crédits de paiement ce programme ça 12 dont doit voir la mise en oeuvre des contrats de plan État Régions et interrégions pour 2021 2027 des des CPE et leur volet territorial, je veux rappeler ici l'importance de ce contrat, qui doivent s'inscrire dans une logique ascendante de partenariat. De dialogue entre les collectivités locales et l'État, et aussi de décentralisation évidemment qui doivent traduire une stratégie globale d'aménagement et non une addition de projet 28 milliards d'euros de crédits d'État ont été contractualisé dans les CPER L C P I E R pour la 7ème génération de contrat dans un peu moins de milliards pour le volet territoriale, un mot sur le contexte, elle aime pas à craindre pour les dépenses d'investissement des collectivités locales, dernièrement, les magistrats financiers. Prévoyait que la situation la fin de l'année, ne serait pas certainement pas meilleur qu'un demi vingt-et-un or, depuis quelques mois, quelques semaines, les collectivités navigue à vue, songez qu'au début du mois d'octobre, Bercy estimé dans une note confidentielle rendue publique depuis que l'année 2022 s'achèvera sans difficulté pour les collectivités et envisageait même des perspectives favorables pour 2023 permettant de faire face à l'inflation, 3 semaines plus tard, la Cour des comptes est loin d'être aussi affirmatif reste plus plutôt prudent devant les certitudes de lié à la conjoncture économique actuelle dans son rapport, dernier le rap, le la juridiction de la rue Cambon révèle la dégradation rapide de la situation en raison ben évidemment de l'inflation des coûts de service et et des biens de la difficulté de mettre en oeuvre des projets d'investissement, et aussi, traduction de ce problème de les multiplications ces problèmes de l'aggravation des appels d'offres infructueux, ses contraintes s'ajoutent aux inéluctables dépenses contraintes telles que le point d'indice, la revolver des des catégories C ou les rénovations énergétiques auxquels sont confrontés les collectivités locales, dans ce contexte, vous y on comprend bien et on mesure aujourd'hui sur le terrain, combien cela complique fortement la capacité des collectivités locales à lancer des opérations d'investissement, un mot sur la une, c'était également sur les les ZRR les crédits inscrits dans le budget 23 stables pour la haine mais notre rapporteur a indiqué les difficultés financières de celle-ci pour financer les cinq peu, dépenses de fonctionnement et sa difficulté à financer les missions qui sont confiées au fil de l'eau par l'État et pour intervenir à la demande de ses partenaires. Notre rapporteur note également au passage le manque de coopération entre les différents opérateurs partenaires que sont le CEREMA, l'agence la rue l'Anaes, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie et la Caisse des dépôts et consignations, par le biais des conventions la révision programmée de ces conventions qui arrive à terme, devrait être l'occasion justement de rechercher une meilleure cohérence, comme nous l'avions craint ici même lors de la discussion sur la création de la haine, c'était cet établissement public, manque d'une stratégie globale construite avec les opérateurs et souffrant d'une réelle visibilité combien d'élus encore ignore même son existence et ou ou ou une partie de ses missions, autre sujet, la maison des freins service qui est aujourd'hui en phase de stabilisation, les objectifs initiaux de ce point de vue ont été relativement atteint, que ce soit en termes de son maillage territorial, je note que lorsque justement la logique à s'entendre et respecter le résultat est plutôt satisfaisant globalement 2600 structure labellisé à ce jour dans les 2 tiers à l'initiative des collectivités locales constitue une offre réel de services de proximité, oh, elle s'ajoute quand même les 127 buts France service à ce jour, qui doivent traduire véritablement la volonté de l'état d'aller au devant des administrés dans les coins les plus éloignés des services et vers ceux qui n'ont pas basculé vers le digital, trop souvent présentée comme la panacée et une évidence nous pouvons ainsi aussi nous inspirer du rapporteur Delcros sur le financement des réseaux France, service, je pense que ce sera une occasion d'en parler, un dernier mot sur la remise à l'pas des zonages et sur l'attractivité au développement rural, je pense qu'à la dynamisation du dispositif des ZRR pour toutes ces raisons, Monsieur le Ministre, nous nous abstiendrons sur cette mission. Merci, cher collègue, la parole est à madame Martine Filleul, pour le groupe socialiste, écologiste et républicain pour quatre minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, à l'heure de l'urgence du changement climatique et des lourdes contraintes qui pèsent sur les finances des collectivités, nous nous interrogeons sur la vision du gouvernement en matière de politique d'aménagement en effet la politique des territoires est à reconstruire, pour fonder les bases de nouvelles solidarités territoriales, mettre en place des financements pérennes et mieux associer les élus et les populations dans les choix politiques et structurant qui engage l'avenir de leur territoire, les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer pour répondre à ces enjeux, et en particulier ceux de la transition écologique et offrir des opportunités et perspectives nouvelles aux citoyens, chacun doit pouvoir s'y retrouver pour cela, elles ont besoin d'une plus grande autonomie d'action, de mettre en place des stratégies territoriales de déployer des actions d'animation des acteurs de leur territoire, d'organiser le débat avec les habitants, or le chemin qui est pris n'est pas le bon entre les injonctions contradictoires, le passage en force, la pression sur les finances locales, les collectivités perdent leurs moyens et de ce fait, leur pouvoir d'agir, je prends pour exemple Lausanne qui est éloquent : en l'état, c'est un objectif contraignant non concertée, sans outil pour le mettre en oeuvre, laissant les collectivités démunies et suscitant l'incompréhension des populations, or les moyens de la haine cité dédiée au soutien des collectivités territoriales et à leur accompagnement en matière d'ingénierie n'ont pas évolué depuis sa création, l'indicateur du programme relatif au soutien des collectivités en demande d'ingénierie fait apparaître une cible de 500 projets en 2023 accompagné en propre et sur mesure par des services au programme de la haine c'était et 250 projets impliquant un prestataire issus du contrat cadre d'ingénierie ce nombre paraît vraiment bien faible en regard des 25000 communes de moins de 1000 habitants potentiellement concernés, le constat est le même pour les programmes Action coeur de ville ou Petites Villes de demain, par ailleurs, les services publics axes structurants de l'aménagement du du territoire se doivent de répondre à la forte demande des habitants des territoires ruraux, mais aussi de certains territoires urbains, or leur accès leur accessibilité et percuté de plein fouet par la dématérialisation de ses services publics, 14 millions de Français sont touchés par l'illectronisme et un Français sur 2 n'est pas à l'aise avec le numérique, sans compter ceux qui n'ont pas accès à Internet et au matériel nécessaire déjà en 2020 la défenseure des droits dénoncer cette fracture numérique est recommandé de maintenir une alternative humaine au tout numérique car la dématérialisation accélérée des services publics alimentent le malaise démocratique et le sentiment d'abandon, les espaces France services sont encore bien loin de répondre à cette attente, je conclurai donc en disant que, décidément, la politique d'aménagement proposé n'est pas à la hauteur de cette période, aux anges, tant de transition écologique que de justice territoriale. Je vous remercie, merci, cher collègue, la parole est à monsieur Jean-Claude Angela pour le groupe Les Républicains pour quatre minutes.

madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, le budget de la mission cohésion des territoires et ses différents programmes programme comporte des insuffisances certaines ce dont, dont des ce qu'ont déjà souligné les rapporteurs, dont je salue le travail, je ne suis pas loin de partager le constat sévère des associations d'élus concernant ce budget qui rêvait qui révèle un manque de cohérence et de vision du gouvernement concernant la politique des territoires. Le point le plus symptomatique de cette situation et cela a été rappelé, et certainement le budget de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui est très largement insuffisant au regard de ses missions, c'était devrait être l'acteur essentiel de la décentralisation, avec des solutions sur mesure du coup humain adapté à la diversité des territoires, mais ses moyens de fonctionnement sont sont limités, en effet, ce budget ne semble pas prendre en compte l'augmentation des nombreux programmes piloté par l'agence parmi lesquelles Action coeur de ville, territoires d'industrie, petite ville demain ni la montée en puissance de ce programmes

comment justifier que les moyens alloués au programme offrant ce service qui servent à combler la disparition des services publics dans de trop nombreux trucs lampes au territoire soit largement en dessous de ce que préconise l'inspection générale de l'administration, dans son rapport de juin 2021 est encore une fois aux collectivités de compenser les carences de l'État, il n'en reste pas moins que sur le moi, la première maison France : ce service reste la mairie dans chaque commune, plus largement, ce budget a de quoi renforcer l'inquiétude des élus des territoires ruraux en particulier qui ne font part de leur incompréhension relative à la mise en oeuvre de politiques publiques bien souvent mené sans eux, je pense à ce qui a été fait dans le passé dans la loi MAPTAM dans la loi, notre et au renversement de la taxe aménagement et maintenant à l'application Dusan. Je partage d'ailleurs le réquisitoire que nous a livrée et Stéphane Sautarel tout à l'heure pour les zones rurales pour les zones de montagne et pour l'agriculture

indépendamment du niveau d'ouverture de crédits dont je note qu'ils n'ont qu'il augmente pas malgré l'inflation je rappelle au gouvernement que les collectivités n'ont pas besoin d'injonction particulière écologique en 2023 pour présenter les projets vertueux adaptées à leur territoire, le gouvernement et l'État doivent faire confiance aux élus locaux. L'inquiétude réelle, elle résulte certainement d'une forme d'incompréhension entre les élus locaux et le gouvernement, comme l'a montré encore l'absence de discours du président de la République à la tribune de l'association des maires de France, lors du congrès la semaine dernière. Ce budget ne permet pas non plus de dissiper les inquiétudes sur le dispositif des zones de revitalisation rurale que nous souhaitons voir se poursuivre ce dispositif a montré son efficacité et le Sénat bien sûr devra être associé à son éventuelle réforme il ne donne pas non plus le visibilité sur la poursuite, l'agenda rural, même si nous à volonté le travail engagé et qui a rappelé, dans ce qu'on relègue Bernard Delcros ce budget traduit une période de flottement pour la ruralité, alors qu'il aurait pu révéler enfin la vision du gouvernement à court ou à long terme la cohésion des territoires nécessite une prise en compte des spécificités pour forger une armature territoriale de proximité, fondée sur la commune avec des élus qui peuvent réellement compétence. Enfin, mes doutes concerne le budget, ce budget sont renforcés par le contexte économique actuel, donc finalement est donc terminée est-ce que la cohésion des territoires qu'est-ce

Madame la présidente, madame, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la cohésion des territoires est un noble dessein il repose sur la certitude que l'immense diversité de ce qui fait la France et la force de notre pays, cette ambition engage l'État à faire confiance à l'échelon local, ces élus et des acteurs de terrain, elle engage également l'état à leur donner les moyens nécessaires pour agir, des crédits du volet cohésion des territoires du PLF 2023 bénéficient de 17,9 milliards d'euros, dont 329 millions d'euros destinés à la politique des territoires c'est considérable parmi les différents programmes de la mission, l'Agence nationale de cohésion territoriale apporte un soutien en ingénierie aux collectivités et les accompagne dans le déploiement de leurs projets de territoire depuis sa création, notre groupe souligne la pertinence de cet outil au service des élus locaux, en particulier dans les territoires ruraux le PLF pour 2023 attribue à la une, c'était une dotation équivalente à celle des années précédentes, on parle de 20 millions d'euros au titre du budget ingénierie pourtant la une, c'était a atteint la plupart de ses objectifs et son cahier des charges a été progressivement élargi, il est dommage que ce PLF n'ajuste pas les dotations de la haine, c'était à l'ampleur de ces missions, les prochains mois seront je l'espère, l'occasion d'engager une réflexion sur le futur de cette agence, je salue la poursuite des politiques ambitieuses en faveur des petites villes et des espaces ruraux le programme Petites Villes de demain, par exemple, permet à 1600 commune de bénéficier de moyens supplémentaires, ce sont les élus eux-mêmes, qui définissent leurs priorités qui pilote leur projet, c'est une bonne approche qui permettent aux habitants d'être mobilisés au même titre que les entreprises, les élus, les professionnels et l'ensemble des acteurs du territoire près de 2200 espace France service My l'ensemble du territoire national et permettent de maintenir une offre de services publics de proximité, ces maisons aide réellement les Français jusque dans les territoires les moins facile d'accès, grâce à des bus itinérant le PLF leur consacrent 36,3 millions d'euros pour 2023, c'est une bonne nouvelle car cette politique a du sens, en revanche, si nous voulons que les politiques en faveur de l'attractivité des territoires ruraux soit couronnée de succès, il faut résorber les zones blanches en matière de numérique et de réseaux mobiles les conseillers numériques France service accompagne accomplissent un formidable travail au quotidien, c'est un point à souligner, mais cela n'est pas suffisant : les élus locaux, dont nous sommes les porte-voix nous sollicitent régulièrement en ce sens, chacun doit avoir accès à un réseau 4 G et à une connexion Internet de qualité car c'est une condition essentielle au développement de nos territoires, l'État doit être mobilisés pour endiguer les fractures d'usages numériques et d'accès au réseau. Nous pourrons d'ailleurs nous interroger sur les dotations dont dispose la une société en la matière, comme le souhaitait ma collègue, le sénateur vanitas pas lui gagent trop du territoire reste encore aujourd'hui à l'écart des différents dispositifs concernant la politique en faveur de l'hébergement et l'accès au logement, notre groupe s'inquiète des tensions sur les prix, nous appelons également à intensifier les efforts en matière de rénovation thermique du parc immobilier existant le contexte inflationniste, souligne l'urgence des dispositifs en matière de lutte contre la précarité énergétique nous serons attentifs à la mise en oeuvre opérationnelle du Fonds Vert et à sa distribution au sujet de la politique de la ville, les crédits sont annoncés à hauteur de 600 millions d'euros environ, je salue la hausse du budget car les chantiers sont importants, nous pouvons toutefois nous inquiéter de la baisse des moyens relatifs à l'éducation, dans les quartiers de la politique de la ville, l'État ne doit pas laisser faiblir son à son ambition en la matière. Enfin, la poursuite du programme Action coeur de ville va dans le bon sens, tant il apporte des solutions aux défis de la revitalisation et du verdissement des villes moyennes, l'État doit s'appuyer sur les territoires ruraux comme urbains qui sont des moteurs en matière de transition écologique la relation partenariale qui s'incarne notamment par la contractualisation dans les contrats de plan État Région va dans le bon sens, le groupe, les indépendants, accueille favorablement ces crédits cohésion des territoires tout en appelant à poursuivre les dispositifs de soutien en faveur de l'échelon local, les élus connaissent leur territoire, ses enjeux, ses habitants, ils sont en mesure de concrétiser l'alliance de l'écologie et du développement économique local. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement, et pour quinze minutes. Madame Madame la présidente, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les les sénateurs. Je suis heureux de présenter la mission cohésion des territoires dans le cadre du projet de loi de finances pour 2023. Et je commencerai par vous parlez de la politique du logement. Cette politique du logement ne doit bien sûr pas minimiser les difficultés du secteur : difficulté de la demande avec l'enjeu de solvabilité des, des, des ménages, l'accès au crédit difficultés liées à l'offre, alors qu'existent d'importants frein à la construction. Face à cela, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. à travers ce budget ma priorité, c'est d'abord le parcours résidentiel. Ce parcours résidentiel concerne d'abord ceux qui n'ont pas de logement. Le mal logement et le sans-abrisme sont des fléaux contre lesquels nous luttons tous les jours avec des résultats. La politique d'hébergement et d'accès au logement des personnes sans abri ou mal logées, soutenus par le programme 177 vise à permettre l'accès aux logements tout en garantissant une réponse aux situations d'urgence. Le parc d'hébergement, financé par l'État a atteint un niveau inédit de plus de 203000 places ouvertes en 2021, dans le contexte. De la crise sanitaire en 2023, à l'issue d'échanges fructueux avec les associations, les préfectures et les parlementaires. Ayant abouti à un amendement à l'Assemblée nationale, les capacités d'accueil du parc seront maintenus à un niveau élevé d'environ 197000 places. Le projet de loi de finances donne pour cela le programme 177 à hauteur de 2 8 milliards d'euros, un niveau jamais atteint et je peux vous assurer, Mesdames et messieurs les sénateurs, que l'État agit et l'État est très réceptif. Au-delà de l'hébergement d'urgence, la priorité est d'offrir une solution de logement pérenne à chacun le plan logement d'abord initié par le président de la République, il y a 5 ans. Avec ce plan, ce sont 400000 personnes qui ont pu accéder à un logement de passer de la rue un toi. Nous poursuivons nos efforts avec un nouveau plan logement d'abord. 44 millions d'euros supplémentaires y seront consacrés dès 2023. Défendre le parcours résidentiel, c'est permettre à chacun, selon sa situation d'accéder à un logement décent et d'ici, maintenir durablement. Le programme 109 aide à l'accès au logement, finance, les aides accordées aux personnes en difficulté en 2023, ce programme est doté de 13 4 milliards d'euros. On est dans les ménages aux ressources modestes et en les accompagnant dans leurs démarches, ce programme participe à la mise en oeuvre du droit au logement prévue par la loi Dalo de 2007, toujours au bénéfice du parcours résidentiel ma mission et aussi de celle de construire plus et construire mieux. Le programme 135 porte à cette fin, la stratégie gouvernementale en matière de politique du logement et d'aménagement, cette stratégie repose sur les piliers suivants. Et. Construire mieux et moins cher, en accélérant le rythme de construction, notamment en zone tendue en simplifiant l'acte de construire. Accélérer la rénovation et améliorer le niveau de performance énergétique des logements. Avec la politique de sobriété énergétique dans le logement avec le calendrier d'éradication des passoires thermiques et avec MaPrimeRénov', nous avons fait sauter un premier verrou en installant la culture écologique, la culture de l'éco-gestes dans les foyers. C'est un premier acquis précieux et beaucoup d'entre vous l'ont souligné tout au long de nos premiers échanges mais soyons lucides la rénovation thermique n'en est si j'ose dire, qu'à son âge adolescent ce quinquennat doit nous permettre de passer à l'âge adulte, passer du mono geste à la rénovation performante, passer de l'individuel au collectif, passer de la structuration d'une filière naissante à la consolidation d'une filière puissante et nous nous en donnons les moyens. Le PLF 2023 prévoit de 45 milliards d'euros sur le dispositif MaPrimeRénov'financé par le programme 174 qui sera discuté cet après-midi et un renforcement sur le programme 135 des moyens de Lana en faveur notamment de la rénovation énergétique pour consolider la dynamique inédite lancée dans la relance. Notre accélération se traduira par un meilleur accompagnement des ménages à travers le service public France rénovent par la poursuite du soutien aux copropriétés de tout type, l'aide MaPrimeRénov'co-propriété sera prolongé pour accentuer l'effort de rénovation des logements en collectif et nous travaillerons à l'accompagnement des copropriétés toutes les copropriétés. Un mot. ça a été évoqué aussi, s'agissant de l'adaptation des logements au grand âge et de la promesse de campagne du président de la République de lancer ma prime adapte une aide unique, simple et attractive. C'est évidemment l'une de mes priorités et le budget que je défends, doit permettre à l'un quasi-doublement du nombre de logements adaptés, l'année prochaine pour amorcer la dynamique se concrétisera par le lancement de la nouvelle aide en 2024. En matière de logement social, ce projet de loi de finances préserve le modèle de financement du secteur, qui fait face à des objectifs ambition prolongation des avantages fiscaux, la TFPB stabilité de la RLS. La contribution d'Action Logement au FNAP Fonds national d'aide à la Pierre, que vous avez supprimé constitue à mon sens un élément essentiel de cet équilibre. Les discussions se poursuivront, bien sûr, pour renouveler la convention quinquennale et assurer collectivement le bon financement du secteur en parallèle des travaux pour conclure un pacte essentiel de confiance avec l'ensemble des acteurs du logement social. ça a été évoqué aussi mon ministère n'est pas que celui du logement, c'est aussi celui de la ville et des quartiers populaires, la politique de la ville intervient dans 1514 quartiers prioritaires où vivent plus de 5 5 millions de nos concitoyens, elle fédère l'ensemble des acteurs qui est con qui concourent l'État, les collectivités, les associations et bien sûr les habitants, permettez-moi, à ce moment de souligner l'excellent travail du rapport des sénatrice Valérie Létard Dominique Estrosi Sassone et Viviane Artigalas, qui seront un outil très précieux de la réflexion sur les nouveaux contrats de villes. Les crédits de la politique de la ville, regroupés au sein du programme 147 et les Agence nationale pour la rénovation urbaine joue un effet de levier indispensable pour. Réduire les écarts de développement entre les quartiers et les autres territoires et améliorer les conditions de vie des habitants. Pour 2023 la politique de la ville, fait l'objet de nouveaux efforts, ces crédits viennent pérenniser notre action dans les quartiers avec l'opération Quartiers d'été et les autres opérations d'dans d'autres Budgets mes vacances à prenante notamment, qui seront des éléments essentiels dans nos quartiers, dès l'été prochain. Renforcer aussi la présence humaine dans les quartiers avec les adultes relais prolongé comme cela a été indiqué les cités éducatives et comme l'a souligné, Madame la sénatrice avait. Enfin, bien évidemment poursuivre le financement du nouveau programme de renouvellement urbain, au total ce sont 37 2 milliards d'euros de contribution totale des ministères concernés. Nous voulons aller plus loin en apporte en portant l'ambition quartier 2030, par le président de la République, dont les nouveaux contrats de villes seront l'outil et le chemin en donnant la parole aux habitants en reconnaissant leur place dans la République, nous construirons des quartiers qui donne le pouvoir d'en partir, mais surtout l'envie d'y rester. Enfin, la mission porte également les crédits en matière d'impulsion et de coordination de la politique d'aménagement du territoire. Le programme 112 qui représente 262 millions d'euros pour l'année 2023 a pour ambition d'accompagner tous les territoires, dans les grandes transitions et leur donner les moyens afin d'aménagement durable. De notre pays et de lutter efficacement contre les fractures territoriales. Ces crédits en hausse de 6 % par rapport à l'année 2022 concourt à la réalisation de 3 objectifs principaux. Apporter des moyens renforcés à l'Agence nationale de la cohésion des territoires là une c'était afin d'assurer un meilleur appui auprès des collectivités. Accompagné aussi les grandes transformations territoriales au travers du déploiement de programmes d'appui spécifique, ces programmes, vous les connaissez, vous les avez cités se sont France services Petites Villes de demain territoires d'industrie nouveaux lieux nouveaux liens Action, coeur de ville agenda rural ou encore le plan France très haut débit. Enfin inscrire avec l'État dans la durée, grâce au contrat de plan État-Région coopèrent et au contrat de relance de transition écologique, ces nouveaux contrats territoriaux représente une avancée. Car pluriannuels globaux et passé est basé sur une apprend une approche différenciée en fonction des régions. Mesdames et messieurs les sénateurs, ces programmes sont essentiels pour nos concitoyens, pour notre territoire partout sur notre territoire pour ces raisons, je vous invite à voter ces crédits, je vous remercie. Merci, monsieur le Ministre, alors nous allons procéder à l'examen des amendements portant sur les crédits de la mission cohésion des territoires figurant à l'état B. Et de suite, je vais vous redonner la parole monsieur le Ministre pour l'amendement 1218 du gouvernement. Merci madame la la présidente, mesdames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les les sénateurs. Le gouvernement vous propose un amendement important pour abonder les crédits d'un peu plus de 30 millions d'euros pour les métiers de la branche action sanitaire et sociale, conformément aux annonces et de la Première ministre et du ministre des solidarités cet abondement et l'équivalent de la hausse du. Point d'Addis de 3 5 intervenue pour la fonction publique et qu'il est important de faire profiter aussi l'ensemble des métiers de la branche action sanitaire et sociale. Voilà. Très bien l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, alors effectivement il y a beaucoup de métiers, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, centre d'hébergement d'urgence et très nombreuses structures et associations qui participent à mettre en oeuvre une politique publique et paraît approprié pour la, pour la commission de le reconnaître en finançant cette revalorisation précisé par par le ministre sera un avis favorable. Merci, alors je vais mettre aux voix, donc l'amendement du gouvernement qui a reçu un avis favorable de la commission qui est pour, qui est contre qui s'abstient et donc adopté l'amendement 1058 Madame Artigalas Saint-je monsieur Bois-d'. Demande de retrait, merci le 1063 madame Artigalas. Merci madame la présidente, après la crise sanitaire et les ménages modestes sont de nouveau fragilisée par la flambée des prix de l'énergie, cette situation met en lumière à la nécessité d'accélérer la rénovation énergétique en favori priorisant les ménages précaires avec la mise en place d'un zéro reste à charge, il faut favoriser des travaux plus ambitieux pour qu'enfin on on perçoit les signes concrets d'une transition énergétique encore trop inefficace encore trop inégalitaire 3 5 6 millions de foyers, soit près de 18 % de la population sont concernées par la précarité et l'exclusion énergétique en France, rappelons qu'il y a par ailleurs urgence les logements les plus énergivores vont disparaître progressivement du marché de la location pour les logements Seger cette interdiction entre en vigueur au 1er janvier 2000 vers deux 3 or 85 % des chantiers financés par l'Anah concernant encore des opérations mono ne permettant ni de réduire la précarité énergétique, ni d'être efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique, trop peu de personnes s'engage dans un parcours de rénovation globale les raisons en sont simples près de la moitié des ménages résidant en passoire technique thermiques ont des faibles revenus et 62 % ont plus de 60 ans MaPrimeRénov'sérénité là de pour les ménages auraient sur des ressources très modestes et financé par le budget de l'ANA et soutient les rénovations qu'en disant un gain énergétique minimale de 35 notre amendement propose de renforcer cette aide pour réorienter massivement l'action de l'vers les logements classés F ou G via un mec mécanisme d'aide complémentaire qui permet une Ride voici on global et un reste à charge zéro. la la la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, qui est en effet toujours souhaitable de favoriser des rénovations globales toutefois madame la sénatrice, j'ai rencontré la directrice générale de la, de l'qui n'a pas formulé une telle demande de crédits supplémentaires et qui a surtout souligné, je partage ce constat, la difficulté, nous avons face à nous, qui est celle de l'absence d'un véritable écosystème d'entreprise générale capable de réaliser des rénovations globales pour le parc privé, c'est aussi la difficulté pour les particuliers d'organiser de tels travaux, en tant que que que maître d'ouvrage, donc, à ce stade de notre histoire, c'est une un avis de retrait sinon défavorable. madame la sénatrice, vous avez raison, la rénovation thermique de l'habitat individuel comme de l'habitat collectif est une priorité que que nous partageons MaPrimeRénov'sérénité, donc la partie qui aide les ménages, les les plus modestes et tu as a déjà atteint un budget de. Plus de 500 millions d'euros, il a été augmenté en 2023 de 130 millions d'euros dans le cadre des aides préalables, plus de 80 % des ménages qui ont été aidés par ma prime sont des ménages modestes mais comme ça a été dit par monsieur le président, à ce stade, la filière n'est pas prête et, surtout, le nombre de dossiers qui arriveraient ne correspondrait pas à une augmentation aussi importante de de cette demande, je peux vous assurer de notre mobilisation, la mobilisation de l'ensemble des des services celle de de l'pour accompagner la demande pour accompagner tout à la fois les ménages les plus en difficulté, qu'il soit en copropriété où on est en habitat individuel mais à ce stade, nous vous proposons plutôt un retrait sinon ça sera un avis défavorable car cette augmentation d'autant plus gager sur le 177 ne nous paraît pas opportun. Merci, merci Madame Lienemann. Notre groupe soutiendra l'amendement de du groupe socialiste et de Madame Artigalas pourquoi, bien sûr, en l'état actuel, on va pas brutalement, pouvoir faire 0 charge 0 reste à charge surtout ceux dont on aurait besoin de d'engager pour atteindre l'éradication des passoires thermiques néanmoins la de la de réhabilitation globale pour ces ménages là est une question centrale, donc il serait quand même important qu'on puisse au moins à titre expérimental sur un nombre par exemple limiter contingentées d'opérations de tester l'idée du zéro reste à charge avec un complément de Lana parce que si cette méthode marche, ça prouve bien que on n'atteindra pas les objectifs de la loi climat-énergie sans ce travail majeur sur le reste à charge des familles modestes et fermé d'un d'un revers de main l'opportunité de commencer à s'engager dans cette voie, nous paraît une erreur, alors oui, la filière, il y a un problème, enfin, on va attendre combien de temps, d'avoir résolu le problème de la filière, alors qu'on a des exigences qui sont fixées par la loi à du délai maintenant rapide et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire s'il y y a pas d'obligation de faire des travaux, il y a pas assez de travaux pour développer la filière et si la filière n'est pas suffisant, on dit qu'on ne peut pas faire des travaux, donc nous soutiendrons cet amendement. Merci madame Artigalas. Oui je je vais retirer cet amendement parce que, effectivement, la ligne budgétaire sur lequel on prend les crédits ne me paraît pas être voilà mais c'est vraiment un demande d'appel je crois que Madame Lienemann a raison : on est vraiment dans une situation où des logements vont sortir du marché très rapidement et puis des personnes qui sont en précarité énergétique, il faut vraiment travailler à ce 0 reste à charge et bien évidemment à aussi à la réorganisation de la filière, je suis d'accord avec le avec le rapporteur mais je bon je le retire, mais vraiment, c'est un sujet qu'il faut absolument regarder de très très près et très rapidement. Merci, cher collègue, l'amendement 1082 Madame Lienemann.

un avis de de retrait ou ou défavorables, comme le rapporteur. Merci Madame Lienemann. Cet amendement concrétise ce que j'ai expliqué en en déclaration générale à savoir quand même la faiblesse du forfait charges or sait qu'hélas ses dépenses de chauffage et de charges vont continuer à peser lourdement s'il a pas dès cette année une amélioration de ce forfait au-delà des deux euros on va durablement et dans un décalage entre l'évolution des APL, est ce que les foyers doivent payer dans leur quittance, donc nous avons proposé un une un abonnement de 500 millions pour ce ce chapitre, je rappelle à 1000000 un milliard cinq tous les ans, économiser par la mise en oeuvre de la compte contemporanéité, donc on a pénalisé les plus pauvres pour alors que là, on aurait pu au moins redistribuer cette somme. Alors je mets aux voix l'amendement 1082 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté, Madame Lienemann pour le 1084.

nous sommes défavorables à la RLS, je rappelle que la Cour des comptes avait fait un rapport montrant que l'instauration d'fragilisé dans la durée, les capacités des organismes HLM à construire et à rénover

Madame la présidente, il se trouve que un nouveau pacte de confiance doivent être négociées dans les, dans les mois à venir entre les acteurs du du logement, il est trop tôt pour que la loi intervienne d'autant que le problème n'est pas immédiat, les organismes de logement social sont dans leur grande majorité, dans une situation saine et l'enjeu est de faire en sorte qu'il puisse continuer à investir à rénover leur parc dans les années et décennies à venir. Je suis très. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Madame la présidente, madame la la la, sénatrice-vous votre amendement évoque une baisse de la RLS, comme ça vient d'être dit par monsieur le rapporteur, c'est ce sont des débats qui doivent être engagées dans le cas de, de, d'une réflexion plus large sur le financement du logement social et hé hé bien évidemment dans le cadre du pacte de confiance en en l'état des choses, moi je, je crois qu'il faut bien évidemment continuer à financer le FNAP dans la situation actuelle, le financement, telle qu'il est proposé par Action Logement correspond à un état des échanges que que nous avons avec eux et, et, de toute façon, pour ma part la la proposition qui avait été celle-là. Sur le logement, qui était un basculement un vase communicant entre le financement du FNAP par Action logement en faisant financer le FNAP par les bailleurs n'était pas la bonne solution, donc il faut continuer à échanger aujourd'hui et les capacités manière, j'aimerais beaucoup qu'on dépense la totalité de de l'argent, inscrite au Fnac qui montrerait la la réelle dit dynamique que l'on aurait partout pour construire plus de logements malheureusement depuis quelques années, la totalité de l'argent, inscrit au FNAP n'a pas été dépensé, donc, à ce stade, je vous propose ou un retrait ou un avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre, Madame Lienemann. je rappelle qu'il y a un décalage souvent entre les orientations données par l'État, qui privilégie la réalisation de PLS et la mobilisation du FNAP

mais je partage votre point de vue, Monsieur le Ministre, l'argent doit être dépensé ça sert à rien de laisser dans les caisses pour des journaux meilleur espère néanmoins votre argumentaire monsieur le le rapporteur, que je peux comprendre sur faut attendent le pacte de confiance mais le pacte de confiance il dépendra de ce qu'il y a dans les inscriptions budgétaires parce que, dès cette année, on va avoir un problème d'abord d'abondement de l'aide à la Pierre, dès cette année, notre Sénat devrait donner un signe politique d'une résorption progressive de la RLS qui pénalise les HLM.

de manquer sans doute aussi un amendement d'appel pour dire que le problème est là : il faut revenir sur cette RLS. Merci, alors je mets aux voix, madame la présidente, l'état. Oui, madame la présidente, très brièvement, mais juste pour rejoindre mes deux collègues, même si on sait que c'est un amendement d'appel vu l'affectation des crédits, on est tous bien d'accord, mais c'est vrai que cette RLS, elle pénalise tout additionnant a ça, effectivement, les modalités d'abondement du FNAP qui ne sont pas satisfaisantes parce qu'effectivement dire qu'Action Logement préfère que ce soit les bailleurs qui finance, c'est quand même moyen le à l'origine, elle est quand même abondé par l'État et l'État pourrait prendre sa part dans le financement des politiques du logement mais évidemment qu'il faut revoir la RLS et très, très rapidement, sans attendre l'exercice budgétaire prochain. Merci, alors je mets aux voix donc l'amendement 1084 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre.

Merci madame la présidente, autrement il propose tout simplement de supprimer le mois de Clarins pour l'ouverture des droits au logement à ce délai de carence qui perdent, ils allaient ménage suis s'installe dans un logement sont venus tous s'ajouter toutes les économies budgétaires réalisées depuis 2017 sur les aides au logement, économie, qui représente quand même aujourd'hui plus de 10 milliards d'euros, il nous semble que dans ce contexte actuel de la protection de nos concitoyens les plus fragiles de doit être dit menacé ni même questionner plus de la moitié des bénéficiaires des aides au logement, de travail, des appels ont démontré une réelle efficacité pour aider par exemple un jeune travailleur à s'insérer dans la société, la réduction de la précarité d'accès au travail concerne de stabilité dans le logement, enfin, je rappelle que le principe, c'est ta main et fait l'unanimité en séance dans nos débats sur la proposition de loi de nos collègues en juin 2000 sur l'efficacité de la lettre même amendement et comme vient de le dire, notre collègue, nous l'avions voté la suppression de ce mois de carence à l'unanimité, à l'occasion de la PPL proposé par notre groupe. Merci l'avis de la commission sur ces deux amendements, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, ce sont des amendements qui aurait un coût élevé : 250 millions et d'autre part, il n'est pas sûr que leur mise en oeuvre soir aisés, notamment parce que cela suppose une modification des systèmes d'information et en tout état de cause, il s'agirait de mieux définir les les conditions des des aides qui sont, qui sont versées, telle que l'avait prévu le Sénat en 2020 à travers une proposition de loi qui supprimer ce ce mois de carence. Merci l'avis du gouvernement, chez le ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Monsieur le le sénateur effectivement vous vous proposez de de supprimer le le mois de carence à l'attribution de l'aide au logement d'abord ce mois de carence n'est pas propre au aux APL, c'est une règle permettant. De vérifier dans l'ensemble des des prestations sociales, la, la, la, l'étude du du dossier et éviter des des versements indus ou des des néanmoins, vous le savez, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas ce ce mois de carence lorsqu'il y a un déménagement lorsqu'il y a une personne qui passe d'une résidence sociale à un habitat pérenne pérenne et et dans un certain nombre de cas d'urgence ces ces mesures de de de carence n'existe pas et comme l'a rappelé le rapporteur, à ce stade, cette mesure aurait un coût très important prix gagées sur le programme 177 et donc pour ces raisons, j'émets un avis défavorable. Merci, alors je mets aux voix l'amendement 1062 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

alors 2 amendements en discussion commune le 391 madame mange. Oui merci madame la présidente, selon un rapport de la Fondation des femmes de 2021 titré : où est l'argent pour l'hébergement des femmes victimes de violences, il est noté que souvent pour faire cesser les violences, la seule solution pour les femmes et la décohabitation, or, le rapport note que près de 40 % des femmes victimes de violences, dont un tiers avec enfants qui ont demandé un hébergement n'ont pas obtenu de solution quatre demandes sur 10 n'ont pas été suivie d'une mise à l'abri les spécialistes des associations et des services publics dédiés aux violences sexistes et sexuelles dans le Haut Conseil à l'égalité, estime à un milliard d'euros les moyens nécessaires à la lutte contre les violences faites aux femmes, selon le même rapport de la Fondation des femmes 20000 femmes ont besoin d'un hébergement d'urgence et d'après le rapport d'information de la délégation aux droits des femmes n'ont pas d'ici mais de l'Assemblée nationale sur le PLF le nombre total de places d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales atteindrait aujourd'hui 11 enfin, 11 1000 11 1000 places à la fin 2023 il manque donc 9000 places d'hébergement d'urgence le coût approximatif d'une place en CHRS étant de 18000 euros simple règle de 3, cet amendement se propose d'investir 162 millions d'euros supplémentaires pour qu'il n'y ait plus 4 femmes sur 10 qui demande en vain un abri d'urgence, j'invite tous mes collègues solennellement sur tous les bancs, à voter cet amendement pour réduire un peu le retard de la France dans le combat contre les violences conjugales et qu'on ensuite, puisque nous allons voter, j'espère, j'invite le gouvernement à lever le gage. Merci et le 1000 53 monsieur Gold. Oui merci madame la présidente, dans le même état d'esprit que que l'argumentaire de précédents, nous finissons donc l'année avec 102 féminicides dont une grande partie de femme tuée chez elle un nouveau Pack un Pack, nouveau départ plutôt devrait être expérimenté dès le début de l'année prochaine pour prévenir les faux départ, le domicile en améliorant la prise en charge des victimes et pourrait comprendre une proposition d'hébergement d'urgence, ce n'est pas suffisant nous manque encore de structure donc le présent amendement propose la création de 1000 places dur d'urgent d'en augmentant de 5 millions d'euros les crédits consacrés à cette politique. Merci la avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, il y a déjà une chose que je comprends pas c'est la mécanique ces deux amendements, c'est-à-dire 162 millions pour le 391 pour créer 9000 places et 5 millions pour en créer mille je trouve ce ce coup étonnamment faible mais sinon depuis plusieurs années un contingent spécifique places destinées à des femmes victimes de violences a été identifié dans dans le parc d'hébergement d'urgence et j'ai noté que, selon les documents budgétaires près de 4500 places sont dédiées aux femmes victimes de ces violences dans le parc d'hébergement d'urgence que je viens de de mentionner, et notamment en CHRS et dans certains autres dispositifs 418 places, le dispositif d'aide au logement temporaire ou elle peut être que le ministre-pourra donner des chiffres encore plus précis que ce que je viens de de verser au débat, alors que bon, nous devons, nous, on a, on a un projet de loi de finances pour 2023 qui finance 1000 places supplémentaires sur ces différents dispositifs, donc il faut reconnaître qu'il y a une prise de conscience progressive est-elle à la hauteur de l'histoire, évidemment c'est c'est c'est la question, madame la sénatrice, mais on peut dire aussi que le parc d'hébergement d'urgence n'a pas vocation à traiter tous les cas de femmes victimes de violences qu'est la réponse normale et et quand même l'éviction du conjoint violent afin que la femme puisse rester au domicile conjugal, le parc d'hébergement d'urgence destiné au cas où cette réponse par défaut ne peut pas être apporté immédiatement donc en l'état au bénéfice explication en attendant celle du ministre, ce sera un avis de retrait sinon défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Monsieur le le sénateur bien évidemment la question des des femmes victimes de de violence est une question prioritaire et et vous le savez, du gouvernement précédent, comme de celui-ci, entre 2017 et 2022 c'est 76 % de places supplémentaires qui ont été dédiée aux femmes victimes de violences conjugales et et à leurs enfants,

la première ministre a annoncé lors du 3ème anniversaire, si j'ose dire du du Grenelle des violences faites aux femmes, une augmentation de 1000 places supplémentaires pour atteinte, comme vous l'avez dit madame la sénatrice 11000 places à la fin 2023, c'est donc 110 millions d'euros qui sera consacrée à ce parc dédié et en plus en fonction des besoins, c'est environ 1 virgule 6 millions de nuitées qui ont été financées pendant l'année 2021. Bien évidemment, cette ce drame dépasse largement la question du nombre de places est une priorité, porté par le gouvernement, mais à ce stade, je ne crois pas qu'il se règle à coups de de financement, mais bien de de prise en compte et et de protection des femmes victimes de violences dans le cadre déjà existants déjà existants et de celui de la progression indiqué par la première ministre. Merci madame la présidente, l'État lui défavorable compris. Oui merci madame la présidente, monsieur Ministre, chers collègues, juste en en réaction à ces deux amendements et en lien aussi avec l'amendement qui portait sur le délai de carence, rappelez-vous, il y a quelques semaines de ça nous avons adopté à l'unanimité un une proposition de loi qui visait à l'aide universelle d'urgence pour les femmes et pour toute personne d'ailleurs, victimes de violences conjugales, elle sert à quoi cette PPL elle sert juste à faire en sorte. Que le premier mois, quand une femme victime de violences quitte le domicile, elle va d'abord vers l'hébergement d'urgence, certes elle a besoin qu'il y ait des places disponibles, mais surtout, cette aide, elle vise à faire en sorte que, hé bien dans ce moi qui la sépare de toutes toutes les aides de droit commun qui mettent un mois débloquer, elle n'est pas comme seul choix de retourner au domicile du conjoint violent et donc quand on parle de délai de carence que je voulais dire Monsieur le Ministre, autant il faut préserver des places certes, autant il faut aussi faire en sorte que dans le délai de carence, on fasse en sorte que les femmes victimes de violences ne se retrouvent pas dans une situation d'emprise financière et obligé de retourner chez le l'auteur des violences, faute d'avoir pu avoir dès le 1er jour le bénéfice de l'APL qui peut la mettre en difficulté financière et avoir le résultat que je ne vous évoquez.

à côté effectivement quelques fois du départ du du du conjoint, vous ne la conjointe, mais c'est à 97 % un conjoint qui lui aussi quelques fois peut être amené plus qu'a amener enfin obligé de partir donc il s'agit bien d'une étude des besoins au parc d'une étude des besoins, on ne parle pas de de toutes les solutions, malheureusement, c'est bien au delà que les les qu'il faut financer toutes les solutions,

voilà, sur les quatre femmes qui n'ont pas un hébergement dont un tiers avec avec des enfants et qui donc reste chez elle, parce qu'il n'y a pas de places d'hébergement, il y a combien de féminicides qu'on calcule moins, mois le retard de la France est probant : il faut faire comme l'Espagne, il faut vraiment avoir un plan, une priorité nationale, ça se traduit dans les priorités budgétaires et c'est pas avec un pas, je ne vais pas dire de sénateur, mais Bill places par an, ben non, il ne faut plus, nous avons du retard, donc il faut démultiplier, il faut que ces 4 femmes et une place et et notamment celles qui sont avec enfants encore plus, donc non je je je n'entends pas votre argument, vous progressez, mais pas assez vite. Merci, alors je mets aux voix donc l'amendement 391 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui. Pour. C'est contre.

Merci madame la présidente, cet amendement, Monsieur le Ministre visa augmenté de 95 millions d'euros, les crédits de paiement de l'action 4 rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie du programme 147 politique de la ville, en effet, l'État s'est engagé à contribuer à hauteur de 10 pour 100 du programme national de de renouvellement urbain, le NPNRU, soit 1 virgule 2 milliards d'euros sur 12 milliards d'euros au total au cours du précédent quinquennat il avait promis de verser 200 millions d'euros, seul 92,6 millions d'euros ont été effectivement payé à ANRU rue le solde est d'environ 1,1 milliard d'euros sur les 10 prochaines années, soit un rythme de décaissement moyen de 110 millions d'euros par an dans le PLF pour 2023 seuls 15 millions d'euros sont inscrits le présent amendement vise donc à porter les autorisations d'engagement et les cris de prime en de paiement à 110 millions d'euros lors de mes auditions, il m'a été indiqué qu'un arbitrage aurait été rendue pour 40 pour garantir 300 millions d'euros sur les prochaines années mais qui serait l'essentiel de la charge pour la période finale, soit plus de 800 millions d'euros de 2000 28 à 2031, je rappelle que ce qui n'est pas mis dans les caisses, maintenant dans les Budgets, devra être mis plus tard donc, cette augmentation est formellement engager sur l'action 4 du programme 135 pour assurer la recevabilité de l'amende dedans. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, le je, je comprends fort bien l'intention de de cet amendement et en profite pour saluer la la force l'engagement notre collègue Madame Madame Artigalas sur ces sujets, de quoi s'agit-il, on a un NPNRU qui doit être pourvu de 12 milliards d'euros, dont 8 milliards apportés par action le logement de 8 milliards par les bailleurs sociaux 1 virgule 2 milliards par l'État qui ont logement et les bailleurs sociaux apportent leur contribution chaque année et ce n'est pas le cas de l'état qui jusqu'à présent, puisque les crédits chaque année sur le programme 147 sont symbolique, très symbolique de l'or de 15 millions d'euros chaque année, d'où le fait que je comprenne bien l'intention de de de cet amendement, de mettre en cohérence les actions avec les annonces pour autant, la rue ne fait pas état pour l'instant de difficultés de paiement, il s'agirait pas pour nous de cautionner un abondement de de trésorerie et une ouverture de crédit ne serait donc en tout état de cause nécessaire que si la contribution des autres partenaires diminué en conséquence, j'ai pas information à ce stade de l'histoire, la difficulté n'est pas à court terme, elle réside dans le la stratégie de financement à moyen terme du NPNRU avec ce sujet d'Action Logement qui nous qui nous préoccupent toutes et tous, voir qui nous révolte parfois puisqu'Action Logement et soumis à une pression sans précédent de la part de la et l'État, qui devra en tirer évidemment les conséquences de tout cela, les conséquences de ses propres décisions, je rappelle que le Sénat s'est opposée au principe de ce prélèvement de 300 millions de de d'actions d'Action Logement prévue par l'article 16 c'est que c'est un acte fort, et j'y vois un appel au gouvernement pour qu'il indique enfin quelles priorités il entend tracer en termes de politique de logement, de l'urbanisme, et tout particulièrement en en matière de renouvellement urbain, donc ce sera, en l'état, une proposition de retrait de cet amendement, après bien sûr avoir entendu le le monsieur le Ministre sur ces éléments. L'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, monsieur le rapporteur, madame la sénatrice. ça a été rappelé, et vous connaissez mon mon attachement et mon attention sur le programme de renouvellement urbain et et sur cette très belle en agence qui est ANRU lors du quinquennat précédent le budget de l'ANRU a loué, est passé de 5 10 puis 12 milliards d'euros, ce qui veut dire que dans les années qui viennent, c'est environ 48 milliards d'euros qui seront dépensés en faveur des quartiers populaires et c'est extrêmement important, c'est une dynamique rarement atteinte et qui continuera à changer la vie, dans, dans, dans ces quartiers, sur ces 12 milliards d'euros, oui, effectivement, l'engagement de l'État, c'est 1 virgule 2 milliards d'euros, je peux vous assurer que la trésorerie actuelle de la rue qui est de plus de 1000 millions ne nécessite pas, à ce stade un un effort supplémentaire de l'État, mais comme vous l'avez dit, l'engagement du gouvernement sur ce quinquennat de 300 millions d'euros sera tenu abondé en fonction des besoins et du travail que l'on mènera avec l'ANRU tout au long des échanges, moi, d'une certaine manière, vous savez. Plus les collectivités font plus l'ANRU a besoin de décaisser, mieux c'est, donc je n'ai aucun doute sur la volonté des uns et des autres de faire, j'étais à Marseille pendant 2 jours pour regarder l'avancée des programmes ANRU je le faisais comme président de la rue et je continuerai à le faire comme ministre-là le l'important pour les quartiers populaires, c'est que ces projets se réalisent et plus on demandera à l'ANRU de décaisser, mieux ça sera, merci. Merci, même la présidente Prima. Merci madame la présidente, moi je soutiendrai évidemment l'amendement présenté par notre collègue Viviane Artigalas, puisque c'est un moment de notre commission, je suis sûre que je ferais plaisir à Monsieur le Ministre, j'en suis certaine pour connaître votre engagement sur le NPNRU, je suis sûr que je ferai plaisir à Monsieur le Ministre, qui aujourd'hui à d'autres obligations, et d'autres contraintes, mais je vous prends au mot monsieur le Ministre, plus on dès qu'elle sera vite plus on sera content, plus nos concitoyens seront contents, donc véritablement le signal que la Commission veut envoyer là, c'est un signal d'accélération de ces opérations de de réaménagement et de rénovation urbaine, il faut qu'on donne aux territoires, la possibilité d'aller plus vite et il faut qu'on donne ce signe de l'engagement de l'État, c'est tout l'objet de cet amendement, qui est un amendement pour nous extrêmement symbolique de la volonté de l'état d'aller plus vite sur la rénovation urbaine, je voterai donc cet amendement. Mais Martigues Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur le rapporteur sur le fait qu'effectivement, il ne la rue n'a pas besoin de trésorerie, ce que, en accord avec la présidente de la commission des affaires économiques, je voudrais vraiment alerter sur le fait que il va voir, on va en avoir besoin très rapidement et ce qu'on ne met pas aujourd'hui en crédits de paiement, on n'est pas certain, malgré l'engagement de de Monsieur le Ministre, qu'il il sera plus je crois que c'est un signe important a donné moi je j'ai quelques doutes parfois sur la possibilité, vos vos marges de manoeuvre par rapport à Bercy, Monsieur le Ministre, donc vraiment je crois qu'il est important que cet amendement soit votée très symboliquement pour bien montrer que l'État s'engage, s'engage dans cette voie, sur des longues années que que demande le et ses financements qui vont être absolument nécessaire pour le NPNRU et vous vous y êtes engagé les Thaçi engagé, il faut qu'il respecte ses engagements. Merci, alors je mets aux voix donc la moment 93 qui a reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il est donc adopté alors 3 amendements identiques, le 362 Monsieur Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, alors les 6 amendements qui suit son d'un même sujet font suite à 2 rapports sénatoriaux sur l'état des ponts en France qui faisaient eux-mêmes suite Monsieur le Ministre au dramatique accident du pont de Gênes, en août 2018 alors le sujet est aussi grave, Monsieur le Ministre, parce que d'abord on a un problème de recensement et d'identification des ponts en France qui est propriétaire de quoi vous avez près de 10 pour 100 des ponts et ouvrages qui sont orphelins et donc, et pour ça, qu'il a dans des amendements pour avoir des crédits de paiement pour ce faire ce travail de recensement parce que à un moment donné, on doit savoir quelle collectivité peut potentiellement être en responsabilité, c'est l'état des ponts a beaucoup changé, la plupart ont été faits avant le 20ème siècle c'est au lendemain de la guerre, c'était pas les mêmes sujets de travaux de circulation, ce n'est pas les mêmes sujets de trafic, les tonnages n'étaient pas les mêmes depuis on a fait aussi le constat que évidemment les épaisses, les épisodes de sécheresse et de changement climatique sont venus affaiblir nos ouvrages d'art et affaiblir les ponts et donc on a besoin de travaux en urgence en urgence parce que on voit bien que ce qui a été fait après le plan de relance ne suffit pas, c'est pour ça qu'on vous demande dans les amendements que l'on a voulu, soit au niveau de la Commission, soit avec notre collègue chaise pour effectivement avoir ses crédits de paiement parce que des travaux doivent être faits et puis alors me dites pas Monsieur le Ministre, que je sais, gagé parce que, en plus, là c'est une question de de sécurité, je vous rappelle quand même que c'est 200 à 200 50 1000 ponts et ouvrages d'art concernés en France, qu'on nous parle de 10 pour sans savoir qui est propriétaire que bien souvent on se retrouve aussi avec des ouvrages d'art et des ponts en Mulliez au milieu rural, c'est le cas de tous les anciens ponts des anciennes lignes de de chemin de fer, on est donc face à des collectivités de petite taille ou des collectivités rurales qui n'ont pas les moyens, ni d'ingénierie, ni les moyens financiers d'engager ses ponts de ces travaux, donc c'est pour ça qu'on a besoin en assistance de maîtrise d'ouvrage du CRM a et évidemment besoin de crédits de paiement, c'est l'objet des 6 amendement madame la présidente, qui suivent et qui sont présentés devant vous. Merci donc, vous avez présenté de 388 également monsieur Chevreau, vous, vous savez le 498. Oui merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est un amendement identique mais qui, qui vise effectivement à créer un programme dédié au sein de la mission cohésion des territoires abondé de de 60 millions pour pour soutenir les collectivités locales dans l'entretien et la réparation des ponts, le programme national pont pilotée par par le CEREMA, qui, qui prévoit des cofinancements et donc on a un besoin de de soutien de l'État, et on a une nécessité de sécurité ces ouvrages, on a, on le doit, on doit cette sécurité à nos concitoyens le sens de cet amendement. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, donc, comme ça été rappelé cet amendement prévoit de créer un fonds pour l'entretien et la et là les réparations aux ouvrages d'art, et notamment au pont qui représente une charge importante, notamment dans les plus petites communes, vous, vous l'avez rappelé alors je souscris bien entendu à cette idée, qui est, qui est une bonne idée, c'est un sujet important, alors le le le problème, c'est que cette ce sujet-là ne relèvent pas de la mission cohésion des territoires, puisque pour les ouvrages d'art et on on on est sur la mission Écologie et transport sur le programme 203 et et j'en profite pour rappeler que dans la loi de finances rectificative qu'on a voté il y a quelques jours, en décembre, on a voté un amendement prévoyant d'abonder à 60 millions d'euros, ce programme sur les ouvrages d'art

en 2023 et d'ailleurs on est précisément ciblée, les communes, parce que c'est bien à l'échelle des communes et des plus petites que se pose principalement cette difficulté à la à l'entretien et la restauration des ouvrages d'art, donc c'est une demande de retrait. Merci, il avait du gouvernement Monsieur le ministre. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur comme ça déjà été dit l'État soutient fortement les, les communes propriétaires d'ouvrages d'art et et de ponts. Grâce aux 40 millions d'euros, l'étude pilotée par le CEREMA a déjà permis l'expertise de plus de 40000 ponts et comme ça vient d'être très bien dit par le rapporteur, c'est pas la peine que je le redise c'est une enveloppe de 50 millions d'euros, qui a été prévu dans le programme 203 et et donc je je partage la proposition de retrait. Merci, alors je monsieur, Explications de vote, madame la présidente, monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre je voudrais à mon tour saluer le travail qui a été conduit sur ces bancs, depuis plusieurs années maintenant, que ce soit par nos collègues m'aurait chaises et Dagbert en 2019 ou plus récemment l'excellent rapport conduit par Bruno Belin, qui est sur tous les bureaux des maires de communes rurales et qui s'en inspire très largement je voudrais également en profiter pour saluer le travail du CEREMA qui accompagne les collectivités seraient ma qui est présidé par une sonner Laurianne, Marie-Claude Jarrot, je voudrais insister pour ma part, Monsieur le Ministre parce que mercredi, nous avions une discussion avec votre collègue sur la prise en compte de la voirie communale dans le calcul de la DSR et on nous a expliqué que finalement on pouvait finalement se passer de ce critère-là et je me dis que finalement il y a une certaine continuité dans les réponses des différents Ministre puisque après ne pas avoir pris en compte les routes communales maintenant finalement ce sont les ponts con sur lesquels on on voudrait fermer les yeux, moi je voudrais insister sur le fait qu'effectivement, c'est un vrai sujet de sécurité, c'est un vrai sujet d'attractivité et d'égalité d'accès de nos concitoyens, un certain nombre de services, que ce soit pour les activités, y compris agricoles qui se déroule dans nos territoires ruraux, que ce soit également pour les infirmières, les médecins qui se déplace à domicile, nous avons besoin vraiment de mettre le paquet sur ce sujet et, effectivement, pour compléter ce qui a été dit sur le défaut d'ingénierie souvent ce que l'on vit sur le territoire, c'est que même lorsque c'est l'intercommunalité qui reprend la compétence hé bien lorsqu'ensuite on recherche des cofinancements, c'est très difficile parce que si vous prenez tous les ponts communaux en compétence intercommunale lorsque vous venez ensuite en commission DETR le préfet vous demande de choisir un ou 2 projets par communauté de communes, et donc vous n'avez pas de subventions, sans parler des départements et des régions ou des fonds européens, qui sont parfois peu attentif à ces sujets, donc on a vraiment besoin d'une mobilisation nationale sur le sujet. Merci Monsieur Beulin.

C'est près de 3 milliards d'euros qui sont aujourd'hui nécessaires, dont 150 millions en urgence, donc je crois là monsieur Miss, on ne peut pas passer sur ce sujet-là, qui touche tous les territoires qui va mettre les élus locaux et notamment les élus ruraux dans une vraie difficulté parce que plus le temps passe, plus les choses se dégradent, donc là ce qu'on vous dit qu'il y a une urgence à être mobilisés, c'est que nous le vivons comme ça a été rappelé par notre collègue Fabien Genêt cette réalité sur le terrain, ça nous est remonté par les collectivités par les les agences départementales qui aujourd'hui accompagne les élus donc, là, maintenant il faut qu'on passe vraiment à la décision, faut qu'on rentre dans l'action, le pont de Gênes, il est dans toutes les têtes, ça peut arriver en France prochainement et on pourra pas dire qu'on est qu'on ne savait pas, donc l'amendement sera maintenu, madame la présidente. Merci oui, monsieur le rapporteur. Oui, juste pour préciser que la demande de retrait de la commission n'est pas attaché à un désintérêt pour ce sujet-là et et je mesure ça de très près, dans, dans mon département, les crédits pour les restes réparation entretien des ouvrages d'art relève du programme 203 de la mission Écologie et transport et non pas de la mission du programme 112 et de la mission cohésion des territoires c'est c'est ce qui justifie la demande de retrait. Merci, monsieur le rapporteur, alors je vais mettre aux voix, donc ces trois amendements identiques : 362 388 498 qui ont reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour.

d'accord, donc 361 386 défendu monsieur Chevreau pour le 497 défendu l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur défavorable, merci l'avis du gouvernement, même avis défavorable, merci, je mets aux voix donc ces trois amendements identiques 361 386 497 avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

Qui est contre. Qui s'abstient sont adoptés alors 2 amendements identiques 374 Madame Estrosi Sassone. Sassone. La présidente, monsieur le Ministre, cet amendement vise à rétablir l'APL accession après accession qui a été supprimée par la loi de finances de 2018 sur les logements neufs qui avait été néanmoins maintenue jusqu'au 31 décembre 2019 sur les logements anciens dans les zones détendues puis qui, en 2019 a été de nouveau mis en application, mais uniquement pour l'outre-mer, illustrant ainsi la politique du Stop and Go, qui a été la politique du logement tout au long de la précédente mandature, cet amendement appel accession c'est un amendement que nous portons ici sur tous les bancs du Sénat depuis sa suppression en 2018 parce que nous considérons qu'il s'agit là d'un outil qui est essentielle pour faire redémarrer le parcours résidentiel, vous avez dit vous-même dans votre propos que vous étiez particulièrement attaché et que le parcours résidentiel était l'une de vos priorités, hé bien, commençons par rétablir l'APL accession parce que nous le savons tous aujourd'hui, bon nombre de ménages et plus particulièrement de ménage dans les zones qui sont extrêmement tendues, ne peuvent pas réaliser leur projet de d'accession à la propriété, d'autant plus actuellement avec la hausse des taux d'intérêt et c'est important aussi parce que ça permet de fluidifier le parcours résidentiel, ça permet de augmenter le taux de rotation dans le parc HLM et donc autant de facteurs qui sont de nature par rapport à la crise du logement que nous connaissons mais surtout par rapport à l'aspiration d'un grand nombre de nos concitoyens de pouvoir soit acheter un logement, soit le construire à travers l'APL accession par également des outils comme le bail réel solidaire ou comme le PS là donc je vous demande véritablement d'entendre ce que nous faisons ici et ce que nous demandons chaque année au Sénat de rétablir cette APL accession c'est 50 millions d'euros, monsieur le Ministre des économies budgétaires, c'est pas par là que ça commence et je vous assure ça permettrait à plus de 300000 ménages aujourd'hui de pouvoir formaliser leur projet d'accession à la propriété. Merci Madame Lienemann pour le 1085 Même amendement que celle de notre collègue Estrosi Sassone juste un argument de plus dans le cadre du parcours résidentiel, on voit des familles qui voudraient accéder à la propriété qui ne peuvent pas parce qu'un problème de solvabilité, notamment parce qu'il a pu l'APL accession qui vont toucher l'APL locative dans un logement alors qu'elle pourrait le libérer et par ailleurs on ferait coup double, favoriser l'accession sociale libérer du logement locatif donc cette accession n'est pas ruineuse pour l'État serait un vrai levier au passage, Monsieur le Ministre, notre Sénat a voté la prolongation du PTZ au-delà de l'échéance de fin 2023, c'est très important pour éviter le Stop Angot de Stop and Go dans le l'accession sociale, quelle sera l'attitude du gouvernement par rapport à ce vote. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Mais la présidente, monsieur le ministre, et est chers collègues, ce sera un avis très très favorable. Merci beaucoup, l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, même avis monsieur le Ministre. Madame la sénatrice, mesdames et messieurs les les sénateurs, vous proposez effectivement de de rétablir la l'APL accession à la propriété, cette extension a été prévu depuis 2018, il a en revanche était maintenu en outre-mer, comme vous l'avez rappelé le gouvernement a privilégié quant à lui, d'autres dispositifs que vous connaissez, que vous avez cité le PSL là le PTZ sur lequel nous souhaitons continuer à à travailler le prêt accession sociale et et bien sûr le le PRS. et, vous le savez, j'en ai pas parlé dans mon discours général mais le le le Conseil national de la refondation que nous avons lancé en en début de semaine, doit être le lieu du travail et de la réflexion, la réflexion la plus large possible sans sans aucun a priori et sans aucun interdit et est-ce que je vous propose, c'est de laisser le temps de la réflexion, le temps de la réflexion au parcours résidentiel et à la capacité de répondre aux différentes difficultés des Français d'accéder au logement, à la propriété et et à la location et donc en attendant, le temps de cette réflexion, ce serait un avis défavorable.

on le sait tous, et je remercie le rapporteur de son très très favorable, parce qu'on on a fait il y a pas si longtemps ici un travail considérable pour permettre à plus de familles d'accéder effectivement la propriété, je pense à l'assurance emprunteur lors d'un côté, on fait des efforts et je ne comprends pas la position de monsieur le ministre, qui est de dire : on va attendre, on va regarder, non, il y a, il y a une nécessité absolue et je soutiens complètement cet amendement, je trouve qu'il est vraiment pertinent et il donne vraiment un signal à tant de familles qui ont un besoin effectivement de pouvoir accéder à cette propriété sur le loger. Merci ma ma président Prima. Merci madame la présidente, naturellement je vais soutenir cet amendement et je remercie le rapporteur également de de son avis, monsieur le Ministre, laisser du temps pour la réflexion, mais vous avez dans ce Sénat des personnes qui sont et vous le savez, des grandes, spécialiste du logement, je parle de Dominique, bien sûr, je parle de Marie-Noëlle, je parle de Valérie Létard, je parle de Viviane Artigalas qui projet après projet qui, rapport après rapport, montre l'intérêt et vous-même d'ailleurs de votre discours, vous l'avez dit le parcours résidentiel est un élément structurant de la politique du logement, cet amendement, il coûte rien, il coûte 50 millions d'euros à l'État, rien, rien du tout et c'est un élément déclencheur du parcours résidentiel, c'est un élément qui va libérer du logement social et qui va donner un coup de pouce récurrent sur le monde du logement et et sur la construction, par pitié, Monsieur le Ministre

à lutter un peu contre la partie sud de Bercy et et s'il vous plaît, restaurer la cohérence restaurer de la cohérence dans le parcours résidentiel on votera bien sûr cet amendement. Merci madame la présidente, l'état. Très rapidement pour dire tout simplement : Monsieur le Ministre, que s'il y a bien un sujet sur lequel on a plus besoin de se faire une idée sur la question, c'est bien celui d'un dispositif qui, depuis très longtemps est identifié dans le paysage comme essentielle à la poursuite d'un parcours résidentiel et n'ayant fait en sorte qu'il ne manque aucun maillon à la chaîne, alors, comme ça a été dit brillamment par tous mes collègues, évidemment on va soutenir cet amendement et monsieur le ministre, il a bien encore une fois quelque chose qui ne souffre d'aucun doute sur son efficience les sa nécessité, c'est bien cet outil de l'APL accession alors vous l'avez entendu Monsieur le Ministre, pourquoi être en opposition à quelque chose qui est juste, la voix du bon sens et du terrain. Merci madame Estrosi Sassone. moi je voulais vous avez fait référence, Monsieur le Ministre, au Conseil national de la refondation, je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus importants qui feront l'objet des travaux du Conseil national de la refondation, je pense en particulier et prenez nous homo sur le statut du bailleur privé, là il y a effectivement des raisons de pouvoir, tous ensemble réfléchir et aboutir sur ce que nous réclamons, ici au Sénat depuis aussi à un certain nombre d'années et donc sur d'autres sujets, mais pas sur celui de l'APL accession ne nous dites pas encore comme bon nombre de vos collègues, on va faire un groupe de travail, on va réfléchir, on fera des propositions non tout de suite, rétablissons cet outil cette aide qui est indispensable pour faire en sorte que le parcours résidentiel, qui est aujourd'hui bloqué, voire complètement bloqué dans les territoires qui en ont le plus besoin, hé bien, puisse enfin redémarrer. Merci, alors je vais mettre aux voix, donc ces deux amendements identiques 374045. Qui ont reçu un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient ils sont adoptés

30000 euros par an en moyenne pour ces maisons France service est loin de couvrir les dépenses engagées par les collectivités, en effet, le rapport du Sénat de juillet 2022 évalue leur coût moyen à 110000 euros par an par an et l'État s'était engagé à participer à hauteur de 50 % du coût annuel d'une maison France service dans le cadre du PLFR 2022 Le Sénat a voté un amendement porté par notre collègue Bernard Delcros, qui prévoit une hausse de 12 5 millions d'euros, soit 5000 euros supplémentaires par maison pour 2022, c'est une première étape, mais on reste loin du compte, compte tenu de la situation financière des collectivités qui portent parfois plusieurs maisons France service car majoritairement situés dans des zones rurales peu denses notre amendement propose d'augmenter la participation de l'État de 50 millions d'euros supplémentaires pour 2023 cette augmentation permettra de passer la prise en charge par l'État et ses opérateurs de 30000 à 50000 euros par maison, le déploiement des Maisons France service connaît une montée en charge tant quantitative que qualitative, il est important que l'état il prenne toute sa part, Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. On a la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, ma ma Madame Filleul cet à cet amendement concerne les maisons France service vous savez que c'est un sujet qui me qui me tient à coeur et vous avez fait référence, je, je, je vous en remercie, il propose donc d'abonder les. Crédit France service à hauteur de 50 millions d'euros pour porter à 50000 euros par maison la participation finalement le soutien aux collectivités ou aux autres opérateurs parce qu'il y a aussi d'autres opérateurs qui qui porte des maisons France service alors je veux juste je partage évidemment l'objectif et j'ai proposé ces 50000 euros dans le rapport que j'avais présenté en commission des finances, vous, vous l'avez rappelé, je veux simplement rappeler quelques chiffres la contribution le soutien qui est apporté aux porteurs des maisons France service et notamment aux collectivités qui porte environ les 2 tiers des maisons France service c'est 30000 euros mais sur ces trente mille euros c'est 15000 euros pour l'État et 15000 euros pour les opérateurs, ce qui fait qu'aujourd'hui pour apporter ses 15000 euros otite du FN été sur programme 112 l'État consacre à peu près de 37 millions d'euros, je partage l'objectif de porter à 50000 euros, c'est la proposition que j'avais fait et c'est 50000 euros, je propose qu'il soit pris en charge à parité entre l'État et des opérateurs, comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui supposerait que l'État pour Athènes se 50000 euros par maison qui est tout à fait justifiée, ça supposerait que l'État apporte mille euros supplémentaires par rapport à ce qui est apportée aujourd'hui, c'est-à-dire environ 25 millions d'euros dans le, vous l'avez rappelé dans le la loi de finances rectificative on a franchi un 1er pas en apportant 5000 euros supplémentaires donc 12 millions et demi 12,5 millions d'euros, donc ce qu'il manque aujourd'hui, c'est pour rappeler un peu le les chiffre ce qui manque aujourd'hui en participation de l'État pour atteindre les 50000 euros si on reste sur un système à parité avec les opérateurs, ce serait 12,5 millions d'euros supplémentaires je propose un retrait, sinon ce sera un avis défavorable pour les les les chiffre que je viens de rappeler mais aussi, je veux rappeler qu'en 2023 il y aura le renouvellement de la convention avec les opérateurs et et je pense qu'il est extrêmement important qu'conviennent que dans la participation à 50000 euros, que l'on prévoit même objectif que les opérateurs continuent à à à financer à parité, donc on a fait un 1er pas dans le PLFR je propose que, on atteint de la la la, une renégociation de la convention de 2023 et que les opérateurs pour essayer de les amener sur cet objectif à 50000 euros, ce qui nécessiterait, pour l'État, seulement 5000 euros de plus par maison, c'est-à-dire 12,5 millions d'euros, c'est, raison pour laquelle je propose un retrait ou, à défaut, hein, ça sera un avis défavorable. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente, exactement pour le même même raison que que monsieur le rapporteur, entre les cinq mille euros déjà ajouté et la négociation qui doit avoir lieu très vite pour que chacun prenne sa part et notamment les les opérateurs dans les maisons de France service je je propose un un retrait sinon ça sera un avis défavorable. Merci donc je mets aux voix l'amendement 1060, qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

messieurs les députés, Gérard, le seul et monsieur Bruno Millienne nous ont proposé la création de postes de conseiller mobilité dans les maisons France service donc nous reprenons effectivement cette proposition, aurait pour mission d'apporter conseil à chacune et chacun des habitants en ressentant le besoin sur les solutions alternatives de mobilité existante afin de les connu de tous et toutes et surtout de les optimiser cet amendement a pour but de financer donc des ressources humaines, l'article 40 et l'article 47 de loi organique, loi de finances interdisant parlementaire d'augmenter les crédits, la mesure est gagée sur les crédits de programmes d'urbanistes territoire, amélioration de l'habitat, l'objectif est bien sûr que le gouvernement puisse lever ce gage cette mesure allant dans le bon sens pour améliorer mobilité du quotidien. l'objectif que pour les habitants qui sont concernés par les zones ZFE et puis si, avoir une information, un accompagnement, un guichet en quelque sorte, on est tout à fait d'accord, en revanche, il nous semble que adossé ses conseillers aux Maisons France service n'est sans doute pas le bon ciblage parce que vous avez beaucoup de maison France service notamment en territoires ruraux sur lequel il y a pas du tout de ces ZFE alors aujourd'hui il y a déjà d'ailleurs des communes qui ont mis un guichet pour informer les habitants sur les ZFE, mais, mais, très franchement, créer des postes adossé maison France service je pense, c'est pas le bon ciblage parce que la très grande majorité des Maisons France services sont en dehors, et même très éloignés des zones ZFE donc pour cette raison-là, c'est une demande de retrait. Merci l'avis du gouvernement Monsieur Ministre. Même avis que monsieur le rapporteur. Merci monsieur Schily. Très rapidement, la la proposition hé bien détendre un conseil mobilité à l'ensemble des territoires pas exclusivement aux et des feux. Merci, alors je mets aux voix l'amendement 989 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour.

soit environ 35000 euros par ETP afin d'accompagner le lancement de nouveaux programmes via avenir qui permettrait d'adapter les programmes Action coeur de ville et, petite ville de demain aux villages ruraux et hyper-ruraux ces chefs de projet seraient ainsi mis à disposition des communes et des qu'on mettait de communes rurales et paient rural. la commission, monsieur le rapporteur. dans le cadre de ces de ce programme, village d'avenir qui n'est pas encore mis en place, donc ça me semble un peu prématuré, on a déjà aujourd'hui d'ailleurs, et je pense qu'il faudra d'ailleurs un peu mettre à plat l'ensemble des dispositifs d'aide en ingénierie interne aux collectivités parce que on a les chefs de projet, des petites villes de demain, on a les les volontaires territoriaux, l'administration, on a les chefs de projet Coeur de ville, on a aussi une aide sur fabrique de territoire, on a des chefs de projet ou des chargés de mission sur territoire d'industrie en a les conseillers numériques alors généralement, c'est à l'échelle intercommunale ça pose le problème de l'accompagnement de l'échelon communal, je pense que, de mon point de vue, il faut d'abord qu'on remette un peu de, de l'ordre au remettre à plat, en tous les cas, l'ensemble de ce dispositif pour essayer de, non pas de réduire tout créer de de rentre plus efficace et d'optimiser cet cet accompagnement des des collectivités et pour ce qui est de l'échelon communal, je pense vraiment que ce sujet mérite d'être abordé dans le cadre d'un programme village d'avenir qui, j'espère, verra le jour dans le cadre de l'agenda 2ème deuxième génération mais recruté 800, chef de projet pour aider 800 communes finalement parce que l'ingénierie elle existe au niveau intercommunal, mais pas toujours au niveau communal, ça été rappelé créer 800, chef de projet pour aider des des communes on va cibler quelques communes on va laisser beaucoup de côté, donc, je vous propose de reprendre ce sujet au moment de l'examen d'un programme Village d'avenir, donc c'était une demande de retrait. Merci l'avis du gouvernement, monsieur le ministre.

en destination des des territoires et des collectivités, les les plus rurales, ma collègue Dominique Faure a annoncé. Le travail en permanence sur l'agenda rural et et donc, en attendant que tous ces travaux aboutissent, je suis d'accord avec le rapporteur pour proposer un retrait. retrait. J'retiré monsieur merci alors le 1061 Madame Filleul. Oui, madame la présidente, monsieur le Ministre, la question a été largement développé dans les interventions liminaires, le nombre de communes soutenu en ingénierie par la haine, c'était hors dispositif Action coeur de ville ou Petites Villes de demain reste encore trop faible au regard des 25000 communes de moins de 1000 habitants, pour lesquels les moyens d'ingénierie sont souvent très limité, voire inexistant, le Sénat a lancé une mission pour évaluer la réelle plus-Value de la haine, c'était pour les collectivités territoriales, nous verrons les mesures d'ajustement nécessaires mais, dans cette attente, il y a néanmoins urgence pour les territoires à se préparer aux chantiers structurants que sont la transition écologique, la mise en oeuvre, Dusan ou encore l'accueil de nouvelles populations et de nouvelles activités, d'autant que le contexte n'est pas favorable à la crise énergétique qui s'inscrit dans la durée et le retour de l'inflation s'ajoute l'incertitude sur les ressources des collectivités, la mise en place du fond Vert pourrait pallier ce manque de moyens, mais son objectif exact ne paraît pas encore bien arrêtée : ses modalités de gestion pouvant encore être clarifiée, c'est la raison pour laquelle notre amendement propose d'amplifier l'action de la haine, c'était dans son rôle d'appui dédié aux projets territoriaux des petites communes avec une ingénierie sur mesure des moyens suffisants, c'est en effet la garantie qu'il y aura une équité territoriale en faveur des territoires les plus fragiles, c'est la garantie d'être en mesure de concrétiser les grandes transitions dans les territoires ruraux c'est enfin redonner confiance aux élus pour les développements de leurs projets de territoire notre amendement propose d'augmenter les crédits dédiée à l'ingénierie des petits, des projets, des petites communes à hauteur de 20 millions d'euros. ça va, il va s'inscrire dans la la la la continuité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je je connais vraiment parfaitement la question des difficultés de communes, je suis maire, rester maire très longtemps d'un petit village de 400 habitants les difficultés des communes avec des secrétariat de mairie parfois à temps partiel pour arriver à faire face à toutes les les tâches et et, notamment, et notamment à monter des projets et et à les suivre, donc je mesure sa part parfaitement et c'est vrai, vous le dites d'ailleurs, il y a 25000 communes, vous l'avez évalué à 25000 25 1000 communes petites communes de moins de 1000 habitants qui finalement se trouvent en dehors des programmes existants, petite ville de demain, un coeur de ville et autres, donc il y a un sujet sur l'accompagnement des petites en même temps on ne peut pas mettre un chef de projet dans les 25000 petites communes donc c'est un sujet je, je le connais vraiment parfaitement pour l'avoir vécu en tant que maire d'un d'un d'un petit village. Je pense que, encore une fois, et c'est pas pour renvoyer à plus tard le la la question pas question de cohérence au moment où on est quand même nombreux à être d'accord pour défendre l'idée d'un programme village d'avenir ça veut pas dire qu'il y aura un chef de projet dans toutes les communes, mais en tous les cas, au moment où on est d'accord ou on essaie de, de, de, de convaincre en quelque sorte, Dominique Faure la ministre en charge de la ruralité, de mettre en place ce ce programme village d'avenir, c'est vraiment à ce moment-là qu'il va falloir qu'on regarde comment on peut arriver à aider ces petites communes qui ont vraiment, même pas d'ingénierie, très peu de services et qui en même temps, ont besoin de monter des projets, être accompagné dans un 24 qui est de plus en plus compliqué sur le plan administratif, technique et et autres, on pourrait citer des cas et j'ai, j'en connais par coeur, de, de, de regarder à ce moment-là commun, on peut, mais près de vraiment de manière concrète, pas seulement avec des des sauts mais comme de manière très concrète sur le terrain, aider ces petites communes qui, en effet, se trouvent exclus des dispositifs, des programmes qui sont en cours. Même si l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Même avis que monsieur le rapporteur, qui l'a très bien exprimé. Ah merci, excusez-moi, alors je vais mettre Pardon, retrait ah oui, mais en général je demande pas comme ça, parce que sinon on prend la parole, donc je mets aux voix l'amendement 1061 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient ne pas adopter l'amendement 1049 président Ruquier. Merci ma président suis mis mes chers collègues, cet amendement propose de consacrer 16 millions d'euros à la transformation des contrats de volontariat territoriale administration un contrat de chef de projet afin d'accompagner les besoins à l'ingénierie des territoires ruraux, ce recrutement pérenne des postes sables stable plus expérimentés de chef de projet devrait attirer plus de candidats. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur.

je dois le dire, parfois de façon un peu rapide et dispersé sans forcément être être ce ce soutenue par une une une démarche cohérente avec encore une fois des chargés de projet Coeur de ville, chargée de projet petite de mer, chargé de mission, les volontaires territoriaux en en en administration et beaucoup d'autres d'ailleurs sur le il était prévu d'ouvrir 800 postes de volontaires territoriaux administration il y en a que 200 finalement qui ont été qui ont été demandés et pourvu. Donc je pense que, avant de transformer ces ces VTH en emplois pérennes, je pense qu'il faut vraiment, et ça rejoint les discussions préfère mettre à plat tous ces dispositifs de soutien à l'ingénierie dans les territoires pour essayer d'avoir un un un ensemble et un système qui soit cohérent et efficace parce que pour être efficace, moment il faut que ce soit cohérent complémentaires, donc c'est pour ça que c'est une demande de retrait. Merci la du gouvernement Monsieur le Ministre. madame la présidente, monsieur le le sénateur, vous avez raison, le le programme et as un programme de de grande qualité mais néanmoins, je ne crois pas que transformer les les postes soit d'actualité, et au contraire peut-être aurait un effet négatif sur le programme, telle qu'il existe aujourd'hui, et donc à ce stade, je vous propose, comme monsieur rapporteur un un retrait sinon ça sera un avis défavorable.

Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, on le mesure de plus en plus le Lausanne est, et de loin le le dispositif qui va impacter le plus fortement nos territoires dans les décennies à venir, c'est un enjeu effectivement structurant pour ces territoires mais aucune réponse n'est apportée aujourd'hui par le gouvernement pour accompagner les communes à réussir la mise en application sans entraver et en réalité, leur développement et en permettant l'accueil de populations, donc il faut redonner de des possibilités de développement pour cette auras ruraux tout en respectant l'objectif Dusan que que l'on partage par ailleurs pour les raisons que l'on sait lié notamment à la biodiversité, donc cet amendement propose d'expérimenter une aide aux maires ruraux pour des opérations dédié à la réhabilitation, la rénovation ou l'adaptation de l'habitat, ainsi que les les opérations de reconversion du bâti. Et la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, alors notre collègue Franck Montaugé soulève évidemment un sujet important plus qu'important, Monsieur le Ministre et alors en l'état, c'est un amendement que qui ne semble pas devoir pouvoir être adopté parce que on est a priori nombreux à ne pas être dans une opposition entre l'urbain et le rural, je pense qu'il faudrait par ailleurs définir des seuils, il faut définir la ruralité, le cas échéant, il y a des tas de sujets techniques sur lesquels, évidemment, il faut se prononcer sur lesquels se se prononcera la mission de conjoint de contrôle le 14 décembre je profite pour pour pour le dire, on va faire des propositions, je, je pense, très forte, mais je vois Monsieur le Ministre, dans l'amendement de Monsieur Montaugé un appel à ce que vous preniez la mesure de la situation en ce qui concerne Lausanne vous voyez Lausanne il est disséminés dans tous les amendements il impact la ruralité l'urbain, le périurbain, les grands projets, le logement, le logement social, même l'ANRU, monsieur le Ministre et et il met en fusion tout ce palais, voilà, il faut que vous le sachiez, voilà, de sorte que tous les groupes, toutes les commissions se sont mises d'accord pour que ce cette se mettent en place cette mission conjointe de contrôle et qui va faire des propositions extrêmement forte qui auront vocation à devenir une proposition de loi assez rapidement et on ne dit pas qu'on est contre Lausanne : on dit juste que, on veut des assouplissements des aménagements du délai des moyens de l'ingénierie on eux tout ça, voilà, alors ça va un peu mieux faut faut le dire, il y a un petit peu plus de prise de conscience avec ce ce gouvernement mais maintenant on attend les fameuses preuves d'amour, alors en attendant les preuves d'amour, on va faire le 1er pas dès le 14 décembre voilà donc ce sera un retrait sinon défavorable mais Franck Montaugé il faut le prendre au sérieux la parce que ce qui ce

Vous l'avez compris le sujet de la zéro artificialisation nette est un sujet largement prise en compte par l'ensemble du gouvernement, le président de la République, on a parlé lors de son discours au au maire pendant le pendant mon collègue Christophe Béchu a un certain nombre d'engagements auprès de vous pour continuer à travailler, vous venez de le. Vous venez de de le rappeler, bien évidemment, ce chantier est est en cours pour que tout à la fois on puisse avoir une démarche écologique mais en même temps ne pas brimer les les territoires dans leur volonté de développement de développement en terme de de logement de développement en terme et économique et et comme le la. Si le président de la République et et la première ministre un certain nombre d'évolutions sont déjà dans les têtes, notamment sur des projets nationaux et et la manière dont ils seront dont ils seront regarder la l'échelle Dusan et fait partie des des sujets sur lequel il y a à travailler et toutes les portes sont ouvertes, merci. l'heure. à ce stade c'est retrait ou défavorables. Oui merci madame la présidente à à l'adresse de l'ensemble de mes collègues ici présents et du ministre aussi, moi j'adore les preuves d'amour, je sais pas vous voilà et et là elle tarde quand même à venir, on a effectivement des intentions tout à fait louable et qu'on peut partager mais nord de ça rien quoi, donc voilà, par principe et qu'on te tue l'enjeu de l'importance du sujet, j'ai bien entendu qu'il y avait un travail de fond qui nous serez présenté dans la d'un d'un peu je ne retire pas cet amendement et donc je, je souhaite qu'on puisse le voter merci. Merci, alors je me vois donc l'amendement 1059 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre.

afin de simplifier les aides actuelles par la création d'une aide unique à l'adaptation à la perte d'autonomie, nous souhaitons que ce dispositif concerne également les personnes en situation de handicap et pas seulement aux personnes âgées, notamment de Maryse Carrère donc propose une augmentation de 10 millions de crédit à cette fin pour une prise en charge de l'autonomie plus globale, quelle que soit l'âge où la situation de handicap. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, monsieur le Président Riquier et il nous semble que cet amendement est déjà satisfait donc j'en comprends difficilement le le le l'objet par ailleurs des toutes sortes d'aides plusieurs sortes d'aide j'en citerai quelques-unes, très rapidement, un crédit d'impôt pour les travaux, une prestation de compensation pour le handicap versée par les conseils départementaux un prêt travaux accordée par Action logement pour les travailleurs handicapés,

Il fait référence aux personnes sans domicile stable qui sont écartés de la guerre six effective de l'ensemble de leurs droits en matière de partir social de la moindre démarche administrative de la scolarisation de leurs enfants ou de l'accès à l'emploi, si la loi Dalo du 5 mars 2007 reconnu le droit à la domiciliation quand même droit opposable le nombre d'de domiciliation, a connu une hausse significative et Dier auprès des sommes communaux ou intercommunaux d'action sociale ou bien aussi bien que les organismes agréés, ces derniers sont patients saturé des crédits de 7 millions c'est 5000 euros en 2021 et puis en 2022 ont été alloués à ces organismes mais la non pérennisation des crédits perturbe leur fonctionnement le présent amendement propose donc de consacrer 10 millions d'euros supplémentaires au a seulement des associations notamment des dispositifs de la veille et sociale afin de leur permettre d'assurer l'effectivité du droit à la domiciliation des personnes sans abri ou en situation de mal logement. Si l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, monsieur le président, requiers soulève une vraie question que cette possibilité d'élire domicile auprès d'un CCAS et et d'autres organismes, mais évidemment il y a la question qui suit, c'est celle du financement de ces organismes agréés il ne on ne voit pas de trace de financement dans les documents donc je sollicite l'avis du gouvernement. Merci le Ministre l'avis du gouvernement, donc. Merci madame la présidente, monsieur le le sénateur le leur, le renforcement des des moyens alloués à à la domiciliation et est déjà prévu quittes de la stratégie prévention et lutte contre la la grande pauvreté, vous avez raison, c'est un élément essentiel pour un certain pour un certain nombre de nos concitoyens en en grande fragilité pour ma part le financement de de cette mesure est prévue sur le programme 304 inclusion sociale et protection des personnes, du ministère de la solidarité et de la santé, action 19 stratégie interministériel de prévention et de lutte pauvreté, pardon, à hauteur de 7 2 millions en 2000 22 et 10 millions en 2023 et donc l'amendement est déjà satisfait. Merci, alors Monsieur Ruquier vous retirer votre amendement

Qui est contre. Qui s'abstient n'est pas adopté, monsieur le Président, Ruquier, c'est à vous pour le 1052. Comme l'ont dit à signaler la la nation la cohésion des territoires n'est pas adopté des moyens nécessaires pour effectuer l'accompagnement de proximité auprès des trop nombreuses collectivités rurales et hyper rural qui n'ont pas de moyens amnésie Éric territoriale, un bloc de 20 millions d'euros, qui devaient être affectés au sur mesure est utilisé pour financer en partie les chefs de projet, des petites Villes de demain le présent amendement donc j'déjà Brooks vise à conforter les besoins et en la matière, alors lointain de 10 millions d'euros, cette enveloppe pour la porter à 30 millions d'euros en 2023, il s'agit ainsi de rétablir par des moyens des génériques dédié et renforcer la possibilité effective pour les petites collectivités territoriales, soit de répondre aux appels à projets sont de monter des projets sur mesure, notamment en matière de transition écologique et énergétique, ce renforcement des moyens dédiés permettra d'accroître l'efficacité de la haine c'était et de ragots action plus visible dans les zones rurales, les auteurs de l'amendement souhaite par ailleurs la tenue de permanences régulières de ses ingénieurs territoriaux, notamment dans les. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors, cet amendement est identique aux 1061 que vous ne doit d'abord examiner tout à l'heure avec une somme qui est qui est différente, et donc les arguments que j'ai développé tout à l'heure pour demander un retrait reste évidemment d'actualité pour celui-là. Si l'avis du gouvernement, même avis que monsieur le rapporteur, merci les retirer, merci les retirer l'amendement 1079 Madame Lienemann. chers collègues, que le l'APL versée avec une franchise, c'est-à-dire que compte, les gens ont droit à une aide personnalisée au logement inférieure à 24 euros, il ne la touche pas, heures euros c'est pas une petite somme, en tout cas pour un certain nombre de nos concitoyens, ça fait deux cent quatre-vingt-huit euros par an, donc nous trouvons tout à fait injuste que des droits qui sont reconnus ne soit pas finalement touché par nos concitoyens, nous demandons donc que l'APL soit versée au premier euros. Merci la vue de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, c'est évidemment il y a pas de petites sommes, bien évidemment, mais ce que je souhaite aussi versé aux débats, c'est le fait que cela représenterait une aumône complexité non proportionnée à l'aide, certes très limité et et par ailleurs, des coûts de gestion qu'on qu'on soulève, ça et là, donc en l'état, ce serait un retrait, je propose. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. nos notre analyse le le seuil de non versement a été diminué de, de 15 à à dix euros pour faire suite à

donc, à ce stade, je, je suis favorable à un retrait ou un avis défavorable sur cet amendement, cet amendement L'État, à juste titre s'interroge sur le non recours et quand il y a des droits, bah, l'État s'arrange pour qu'il ne soit pas garantie, vous n'allez pas m'expliquer qu'avec la coupe, la complexité du versement des aides qui bien plus compliqué à mon avis, que ce système de versement quand aider les les les APL sont faibles et puis par ailleurs, rien n'empêcherait l'État de décider d'un cumul et de déverser que trimestriellement ou à un moment où effectivement il y a moins d'actes techniques à opérer, donc je maintiens cet amendement. Merci, alors je mets aux voix l'amendement 1079 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour.

Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, cet amendement concerne les services intégrés de l'accueil et de l'orientation, ce qu'on appelle les SIAO qui sommes nous savons tous des acteurs centraux de la régulation du dispositif d'hébergement et de logement adapté mais qui sont aussi la clé de voûte et la cheville ouvrière de la politique publique de l'État en matière de lutte contre le sans-abrisme et du service public de la rue, au logement, compte tenu des objectifs particulièrement ambitieux, que le gouvernement a au SIAO et de ses missions, qui ne cesse de croître pour l'ensemble des personnes qui travaillent à l'intérieur de ces services, il nous a semblé important que nous puissions à travers cet amendement proposé que tous les personnels des services intégrés d'accueil et d'orientation qui assure la prise en charge des difficultés en grand des puissent pouvoir bénéficier d'une revalorisation de la rémunération du secteur et je pense en particulier aux écoutants du 115 qui sont extrêmement sollicités, qui doit faire appel quotidiennement à la détresse des appelants, qui sont souvent confrontés à un contexte de saturation de l'hébergement qui ne leur permet pas d'apporter des réponses satisfaisantes aux personnes qui font appel au au 115 et pour toutes ces raisons, nous pensons sincèrement que un geste en faveur de ces personnels et plus particulièrement des écoutants du 115 serait particulièrement quant à la revalorisation de leur rémunération. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, pour dire que je m'inscris dans les pas de la sénatrice ça sonne pour dire que les les services intégrés de l'accueil de l'orientation, joue un rôle clé qui ont connu des réformes importantes que leur travail est difficile qu'il appelle une revalorisation, cela peut cela peut s'entend, bien entendu, mais il est à noter aussi que que le taux de réponse étant a priori faible il y a plus d'indicateurs budgétaires qui a été supprimé donc difficulté apprécier tout cela une difficulté donc il peut apparaître comme systémique, au final je comprends l'intention qui est excellente, mais difficile à apprécier, parce qu'on n'a pas d'indicateurs précisément donc je sollicite l'avis du gouvernement. Merci, alors l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, très attendu. madame la présidente, mesdames et messieurs les les sénateurs, madame la sénatrice, vous avez raison les les accueille les services d'accueil et d'orientation, les, les, ce sont des acteurs centraux de la régulation du disque. Positif de de l'hébergement et pour avoir été moi-même un certain nombre de soir les rencontrer et voir la la qualité leur de leur engagement et la difficulté de. De leur travail, je je m'associe à vous dans dans le cette volonté de de les encourager et de reconnaître la l'extrême difficulté, vous le savez dans la dans la continuité du déploiement du du du dispositif logement d'abord, le gouvernement a affirmé par l'instruction du 31 mars 2022 une ambition forte pour laisser les SIAO acteur clé, clé de voûte, comme vous l'avez rappelé du service public de la rue au logement. La première ministre la la dit et et afin de soutenir l'engagement quotidien de ces acteurs de première ligne, le gouvernement souhaite effectivement reconnaître la qualité du travail mené en attribuant une prime aux salariés de ses structures SIAO et donc je je confirme l'annonce de la première ministre avec le versement d'une prime mobiles, les modalités de cette prime doivent encore faire l'objet d'un travail, mais seront présentés sous quelques semaines au plus et feront l'objet d'une rémunération en cours d'année prochaine, avec un passage devant la représentation nationale à cette occasion, dans l'attente et avec cet engagement, je vous propose donc de retirer votre amendement, à défaut, mais l'avis sera défavorable, mais je vous assure que cette prime est en cours de préparation. Merci madame Estrosi Sassone. Non, je ne vais pas retirer cet amendement, d'abord parce qu'on l'a présentée aussi au nom de la commission des affaires économiques et qu'il est largement partagée par l'ensemble des bancs de cet hémicycle, certes, vous nous prenez un engagement ou la première ministre la pris disant qu'il y aura une prime qui va être versé au personnel SIAO, nous pensons considérablement que ce n'est pas une prime qu'il faut leur accorder, mais si on veut véritablement continuer à les accompagner dans ses missions qui sont de plus en plus difficulté difficile et leur montrer que nous sommes aussi à leurs côtés, mais que vous le gouvernement, vous comptez beaucoup sur eux pour mettre en place l'ensemble des missions que vous souhaitez sur l'hébergement, le logement d'abord le service public de la rue, au logement, c'est une revalorisation de leurs salaires et c'est véritablement permettre permettre aussi à ce qu'il y ait demain d'autres personnes qui s'engage sur ces métiers-là parce qu'on risque aussi de craindre qu'il y a une désaffection des personnes sur ce type de métier. Merci, alors je mets aux voix l'amendement 372 qui a donc reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre Qui s'abstient, il est donc adopté le 930 Monsieur le Président Maluret. Merci madame la présidente, cet amendement vise à doubler les moyens consacrés à l'agence nationale de cohésion des territoires afin de soutenir son action dans le cadre de l'action France mobile un New Deal a été conçu, conclu en janvier 2018 d'entre le gouvernement, l'Arcep et les opérateurs mobiles historique pour généraliser la couverture 4 G partout en France après une montée en charge progressive au cours des premières années, cet accord engage les opérateurs à assurer la couverture réseau de 800 sites en zone non ou mal couvertes, or les élus locaux font toujours lui valoir que ce rythme est trop lent en particulier n'a pas été révisés à la hausse depuis la pandémie, alors même que le besoin en couverture réseau des zones rurales n'a jamais été aussi fort, compte tenu de la montée en puissance du télétravail et de la nouvelle attractivité des communes rurales, c'est pourquoi cet amendement propose de doubler les moyens consacrés à la une société afin d'augmenter le rythme de ce déploiement et répondent ainsi à la demande des territoires ruraux qui se sentent mise à l'écart du dispositif France- mobile.

à étudier le gouvernement, la commission des des finances sont d'accord pour qu'on aille un peu plus tard et terminé en fait crédits de la mission alors est-ce que quelqu'un s'oppose, on Non, je ne vois pas donc prolonge alors pas trop long quand même, mais en tout cas on prolonge maintenant, je vais demander l'avis de la commission sur l'amendement 930 Monsieur rapport vise, ça a été dit à doubler les crédits destinés au au New Deal mobile alors en abondant à hauteur de 5,6 millions d'euros, alors certes le déploiement du New Deal, Odile, hé bien piloté par la haine, c'était et par l'Arcep, d'ailleurs, en revanche, je pense que les crédits ne figurent pas sur la maison sur la mission cohésion des territoires et donc j'avoue que je ne connais pas le montant alors si je comprends bien, en toute logique, si en abondance de 5 6 millions je les crédits, ça veut dire que les crédits sont aujourd'hui à peu près à 2,8 millions d'euros, du coup, je connais pas exactement le montant qui est consacré, je pense que ça relève pas de la mission cohésion des territoires du coup peut être le gouvernement Monsieur le Ministre, vous nous en direz un peu plus sur le sujet, c'était en tous les cas, c'est un avis du gouvernement, même si évidemment je partage Abdellatif et que le sujet est extrêmement important. Merci madame la présidente, pour aller vite, juste, c'est le le le New Deal, ces 3 milliards aujourd'hui, donc c'est un investissement extrêmement important mais effectivement sur sur d'autres crédits, donc je je propose ou un retrait ou un avis défavorable. Merci, je mets aux voix non vous retirer d'accord merci beaucoup. Monsieur Christian Brunel, vous vouliez prendre la parole, je crois. Oui, madame la présidente, suite à votre demande alors à la réalité, à la demande du gouvernement, vous avez proposé d'aller un peu plus loin, je crois qu'il faut mettre l'explication de texte, voilà qui va avec un peu plus loin c'est pas 14 heures parce que tout simplement on avait un amendement au rythme actuel, c'est une heure donc, ça veut donc dire que sur des amendements qui aurait peut-être un peu moins de profondeur que d'autres. On irait assez vite et garder sur les amendements qui ont vraiment beaucoup de sens pour garder un peu de temps, voilà pour le reste, présentation lacunaires, on va dire, mais tout le monde a le texte, donc tout va bien et puis ensuite, voilà, pas de pas de doublon, et cetera et on ne reprend pas la parole, enfin et nos rapporteurs et le ministre s'astreignent également à une limiter leur position merci. Merci monsieur le président, alors 2 amendements, donc ils font l'objet d'une discussion commune le 1140 monsieur faire Nick. Oui, madame la présidente, donc un amendement profond est censé mais une présentation néanmoins sommaire, les circonstances l'exigent donc il propose de renforcer l'accompagnement et le conseil en mobilité sur tout le territoire urbain comme rural en d'temps les maisons France, service d'une compétence d'accompagnement et de conseil en mobilité pour l'urbain, j'ai pas besoin d'insister et l'excellent travail de notre collègue Jacques hein sur les mobilités en zone peu dense a établi l'enjeu essentiel dans le rural aussi du conseil en mobilité durable. Merci le 167 Monsieur Béland et défendu merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Encore une fois, on l'a évoqué tout à l'heure, l'idée d'informer les habitants qui sont là ou proches de zones ZFE on est d'accord, en revanche, je pense que le ciblage des maisons France service n'est pas bon, vous avez des départements entiers, qui ont beaucoup de mes enfants, service, c'est pas du tout de à feu et à l'inverse, des zones des dans lequel il y a pas de maison France service donc je pense que le ciblage sur le Maison France service n'est pas de bon ciblage on est d'accord sur l'objectif. Donc retrait défavorable sur les, de l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, même admis que le rapporteur OK, alors je mets aux voix le mille cent quarante, qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient, il n'est pas adopté le 167 est retiré Monsieur Béland. Merci beaucoup, alors l'amendement 95, madame Artigalas. Merci madame la présidente, cet amendement vise à augmenter d'un 1000000 55 1000 euros, les crédits de paiement de l'action hein action territorialisée dispositif spécifique de la politique de la ville du programme 147 cet abonnement pour objectif de renforcer dédié au bataillon de la prévention qui doivent mobiliser en binôme 300 éducateur spécialisé et 300 médiateur adultes relais, or les collectivités peinent à recruter ces éducateurs sur des postes à durée limitée est moins bien rémunérés que ce que les mails, même profil peuvent trouver dans le secteur médico-social qui a bénéficié d'une revalorisation décidée par le gouvernement, le différentiel est ainsi de 183 euros Net par mois et par poste 293 euros, avec les charges, l'abondement permettra de combler cette différence sur une année complète, qui ne doit pas rester à la charge des collectivités, cette augmentation est formellement engagé sur l'action IV du programme 135 pour assurer la Russe bah la dignité de l'amendement. Merci la vie de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, madame article à se poser, de poses une question importante et je sollicite l'avis du gouvernement. Si Monsieur le Ministre votre avis avec sobriété.

concrétisés par le déploiement progressif de 600 médiateur à la fois donc sur des postes d'adultes relais et d'éducateur spécialisé dans une quarantaine de quartier, en particulier dans les quartiers de de reconquête républicaine ce dispositif est toujours en cours, en en phase d'évaluation oui les difficultés existent pour le le recrutement des éducateurs spécialisés des, des, des difficultés de dans le cadre de la formation des difficultés dans le cadre de la pérennisation des postes notamment les pour les éducateurs spécialisés, porté par la prévention spécialisée départemental mais je ne suis pas certain que ça ne soit qu'un qu'un problème financier et et pérenniser et pour recruter ses postes, c'est un métier qui a besoin d'être revalorisé et accompagner à ce stade, je, je, je, ça sera un avis défavorable pour continuer à évaluer ce ce dispositif et et ne pas prendre une mesure unilatérale qui ne sauraient pas être mise en oeuvre. Merci, alors je mets aux voix l'amendement 95 oui. Pour intervenir quand même, je crois que c'est très ces postes sont extrêmement importants sur les territoires et je redis, certes le la rémunération n'est pas la seule, le seul frein au recrutement mais c'est ce que nous ont renvoyé les territoires que nous avons vu, s'il y a des vraiment des difficultés de recrutement parce que c'est un métier qui est peu attractif, comme d'autres, bien sûr, mais nous devons en tenir compte. Merci, je pense que c'est voilà. Merci beaucoup, donc je mets aux voix l'amendement 95 qui a reçu, donc un avis défavorable de la commission du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient est pas adopté 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 65 et défendu. Oui, madame la madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, la loi 3DS dans son article 91 instaure un nouveau critère de recours au titre du droit au logement opposable désormais une personne en situation de handicap logée dans un logement inadapté pour entamer un recours à l'amiable ou en contentieux pour être relogés aussi notre collègue Philippe vous vouliez propose cet amendement qui vise à donner les moyens aux pouvoirs publics de garantir une offre de logement et de mieux recenser l'offre de logements accessibles, je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Ruquier pour le mille sept il est défendu, merci la visite de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, je sollicite l'avis du gouvernement, bon, notamment pour savoir quel est son estimation du coût des conséquences la la la loi 3D 3DS sur le coup des contentieux d'allô. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre, sur ces deux amendements. en 2022 afin de répondre à la problématique du handicap dans le logement, le gouvernement a choisi d'instaurer dans la loi 3DS un nouveau critère de reconnaissance au titre du droit au logement opposable Dalo pour les personnes en situation de handicap logée dans un logement cette mesure va accroître le nombre de recours devant la les commissions en haut une hausse attendue de 10 % pour l'année 2023, le gouvernement a tenu compte de cette hausse dans le PLF 2023 en programmant quatre millions d'euros de crédits supplémentaires dédiés au contentieux Dallo ceux-ci progresse de 35 à 39 millions d'euros au PLF 2023, ce qui représente une augmentation de 11,4 %. Donc à haute à ce titre, les motifs de cet amendement, nous semblent satisfaits et j'aimais donc un avis défavorable.

par notre collègue Louis-Jean de Nicolaï, vise à augmenter d'un 1000000 d'euros, le les montants des financements mobilisés par l'État pour la qualité de l'eau dans la très belle région des des pays de la Loire, que j'ai l'honneur d'être un représentant de cette région, donc je dirais de pouvoir le défendre et j'espère que mon collègue Bruno Belin dont on voudra pas, je vous remercie. Merci, alors l'avis de la commission. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre à l'avis du Gouvernement est défavorable. Alors je mets aux voix l'amendement 360 qui a reçu un avis de sagesse de la commission est défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est donc adopté Madame Jasmin pour le 1064. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre notre amendement a pour objet de une égalité ni l'égalité et de rectifier en quelque sorte une situation qui n'est plus qu'il n'a plus d'objet en quelque sorte la proportion de familles de plus de 6 enfants en outre-mer par rapport à celle de l'Hexagone ne justifie pas les mesures qui sont jusqu'à maintenant prise cet amendement est aussi l'occasion d'évoquer la question du de neige qui ne correspond plus aux réalités vécues sur les territoires, c'est particulièrement probant pour les territoires d'outre-mer, classé en zone géographique, alors que les prix des loyers en outre-mer se rapprochent des prix franciliens justifiant la modification du zonage l'amendement propose d'abonder le crédit du programme 109 à l'accès au logement action yeux hein personnel à hauteur de 1 1000000 d'euros, pour assurer la recevabilité financière de l'amendement cette cet abondant

madame la sénatrice, nous partageons l'objectif de de la mesure proposée puisque effectivement cette mesure de différenciation pour les familles de plus de 6 6 enfants en en outre-mer et dans l'Hexagone ne se justifie plus et et donc un arrêté sera publié dans les prochaines semaines afin de mettre fin à la limite de six enfants dans la prise en compte du calcul des allocations logement en outre-mer, cette mesure, qui relève du domaine réglementaire est en cours de prise en compte, je vous propose de retirer cet amendement. Merci ma ma mère.

pour Saint-Martin pour Saint-Barthélemy ça coûte 852000 euros. Merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Alors cet amendement prévoit un crédit de 800000 euros, un petit peu plus 800 5000 euros pour créer des des chefs de projet, attaché à la à raison de un par région, plus les territoires d'outre-mer, ça être très dis très franchement, je pense qu'il faut renforcer les moyens une c'était mais je pense que la chaîne régionale n'est pas le bon aujourd'hui à une personne identifiée d'ailleurs dans chaque département et je pense qu'il faut renforcer les moyens de haine, c'était à l'échelle départementale parce qu'on reste dans une échelle de proximité avec les territoires avec les élus locaux, c'est la raison pour laquelle la Commission demande un retrait.

ça de permettre le recrutement d'une dizaine d'argent d'architecte conseil et paysagistes, conseiller de l'État mis à disposition gratuitement auprès des collectivités territoriales pour les cours de mission d'expertise en matière d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement du territoire, la droite de j'arrive Héroux. Merci l'avis de la commission de ce rapport. Madame la présidente, sera un retrait sinon défavorable. Merci monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, même avis. Oui, le même à vide dans notre analyse, cet amendement est déjà satisfait. Merci retirez-vous retirez merci madame Conconne pour le 1057. Oui, madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues Greenhalgh, sujet : je n'ai pas profond, il est dramatique, comme vous le savez, les îles de Guadeloupe et de Martinique ont été impactés par le plus dur, le plus méchant des pesticides le chlordécone qui empoisonne à la fois les humains, mais aussi les Terres de ces pays pour au moins 700 ans donc, aujourd'hui, il faut savoir que pour nous servir de l'eau potable et donc dépolluer au robinet, les collectivités font des efforts énormes coûteuse pour, entre autres, assainir l'eau avec des filtres à charbon, c'est le seul moyen qui existe aujourd'hui pour nous permettent d'avoir de l'eau non polluée au robinet cette charge et justement à la charge des collectivités et pourtant le président de la République de manière très singulière et je salue cette reconnaissance a reconnu la responsabilité de l'État dans l'empoisonnement au chlordécone à la Martinique et à la Guadeloupe, donc il me semble cohérent, il me semble juste : il me semble équitable que c'est au pollueur à l'État, qui l'a reconnu, de porter la charge qui est estimé pour cette première année à 400000 euros, des frais de dépollution et en particulier d'achat de filtres à charbon qui permettent d'arrêter de polluer et de porter cancer aux habitants de Guadeloupe et Martinique j'espère en tout cas que il y aura un regard. Attentionné à cet amendement. qui ont été rappelés par knock-out collecteur qui sont tout à fait important et on reviendra pas sur le sur le sujet du coup l'État intervienne à travers le plan encore déconne chlordécone en Martinique et en Guadeloupe et à travers un programme des interventions territoriale de l'État, ce qu'on appelle le le PIT, ce qui est prévu dans le but du projet de budget pour 2023, 2023, ces 4 5 millions d'euros, vous proposez d'augmenter ses crédits à hauteur de 500 400000 euros, si je me trompe pas 400000 euros et donc nous devons un avis favorable à cet amendement, mais je tiens à préciser quand même que, finalement, le Parlement a assez peu de lisibilité pour cette action là pour deux comme pour d'autres actions d'ailleurs du programme d'intervention territoriale de l'État, parce qu'en cours d'année, il y a des transferts en gestion et finalement qui échappe finalement à à la Libye à la visibilité du du parlement et, l'année dernière, en plus de ce qui a été votée dans la loi de finances en 2000 22 et 1 virgule 6 millions de crédits qui auraient été transférés en cours d'année, un avis favorable pour rajouter la somme qui est prévue les 400000 euros au programme le plan chlordécone et c'est vrai que les enjeux sont très importants. Merci l'avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Madame la présidente, madame la sénatrice, vous avez raison, le le sujet du du chlordécone est est un sujet grave, il est une priorité de nos collègues, ministre de l'Outre-mer et et du ministère de la santé, ça a été rappelé un un budget inédit est consacré à la mise en oeuvre du 4ème plan national de lutte contre la pollution par le chlordécone ses 92 millions d'euros entre 2021 et 2027 avec 47 mesures, dont 42 ont déjà été et bien évidemment les crédits du programme 162 ne résume pas mais pas du tout les actions des pouvoirs publics en matière de lutte contre les pollutions par le chlordécone, l'action est bien plus large, avec des mesures sur la santé, l'environnement, l'alimentation, la qualité de l'eau, comme vous l'avez dit, mais dans la mesure où où on est bien au-delà de ce programme 162 l'avis du gouvernement, et est un retrait ou sinon un avis défavorable. Merci Madame Lienemann. Oui, je me la commission et soutenu le l'amendement de notre collègue, vous avez vu que les tribunaux ont arbitré pour considérer que ne pouvait pas juger d'une responsabilité des uns ou des autres pour des raisons de délai et le chef de l'État a dit à juste titre, que l'État était responsable, il faut donc maintenant qu'on soit sûr que cette responsabilité arrive sur le terrain en sonnant et trébuchant et j'approuve donc non seulement l'amendement mais la remarque de notre rapporteur, qui doit nous mettre le Parlement en vigilance totale pour être sûr que les engagements pris soient tenus. Merci madame Jasmin. Oui, je suis oui merci madame la présidente, moi je suis vraiment très heureuse de ça fera que la la commission donné un tel vie et ça me permet également de féliciter de travail de l'Opecst l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques avec notre collègue Catherine Procaccia, qui fait un travail de fond et qui est en cohérence avec ce que vient de proposer ma collègue et Catherine Conconne donc je crois que vraiment, Monsieur le Ministre, même s'il y a un certain nombre d'arguments que vous pouvez évoquer, je crois que la commission a eu raison, raison de soutenir et je félicite également les propos de notre collègue, Madame Lienemann merci. Merci, même Conconne. Oui, dans ma dans ma discussion générale d'hier, je parlais d'attention, vous imaginez bien, Monsieur le Ministre, que le plan chlordécone, je le connais pas au coeur que je participe à toutes les réunions concernant le chlordécone j'approuve les sommes qui ont été mises, j'approuve la démarche je, je, il m'arrive même d'aider le gouvernement à le mettre en oeuvre, parce que pour moi il s'agit pas d'une question politique, il s'agit d'une question humaine, il s'agit de questions de santé il y a aujourd'hui des ouvriers agricoles qui meurent à cause du chlordécone, c'est un drame donc aujourd'hui, il faut marquer des intentions et que des collectivités et à payer la dépollution de l'eau avec des moyens de filtres à charbon, ce n'est pas juste le responsable, le pollueur, celui qui a autorisé la diffusion de ce pesticide violent et et dangereux, doit prendre en compte cette dépense, et nous sommes là, entrée d'examiner une une mission cohésion des territoires les les éléments du plan chlordécone, ce sont des éléments qui sont fléchés et vous imaginez bien qu'avant de porter mon amendement, j'ai fait le taux du plan chlordécone aucune ligne ne prévoient cette dépense de remboursement à la collectivité locale, dont sept s'ce sens que je l'ai déposé parce que moi j'estime que là aussi, l'État doit marquer des intentions extrêmement forte et dire aux collectivités locales, nous avons pollué nous vous aidons à dépolluer. Si, alors je mets aux voix l'amendement 1057 qui a reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour, qui est contre qui s'abstient, il est adopté, Madame Artigalas Alès pour le quatre-vingt-quatorze. Merci madame la présidente, cet amendement vise à augmenter de 200000 euros, les crédits de paiement de l'action, hein, du programme 147 avec pour objectif de relancer l'activité de l'Observatoire national de la politique de la ville placée au sein de la haine, c'était en effet l'ONPV est devenue une coquille vide, il n'a plus de président depuis un an et ses effectifs ont été divisés par 5 depuis son intégration à la une or le besoin d'évaluation de la politique de la ville et centrale, à la fois pour mesurer les effets du NPNRU et ceux des politiques de la ville auprès des populations, il est par exemple nécessaire de créer des cohortes poursuivre les parcours des bénéficiaires dans la durée, dans et en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, cette augmentation est formellement engagé sur l'action IV du programme sera pour assurer la recevabilité de l'amendement. Je vous remercie, merci l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, je souhaiterais savoir pourquoi l'ONPV serait une coquille vide, donc un avis du gouvernement sur le sujet. Merci l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Madame la la présidente, madame la la sénatrice Monsieur le le rapporteur, l'ONPV et est tout sauf une coquille vide, vous savez, elle doit je crois être un scientifique et je suis très attaché aux études et à nos capacités d'évaluation de, de, de la politique de la ville, j'ai fait des propositions pour renommer un nouveau ou une nouvelle présidente à à l'ONPV, on travaillera avec et on travaille déjà avec l'équipe de la haine c'était et et son nouveau directeur, pour que l'ONPV mais j'ai rencontré les équipes actuelles, donc c'est pour ça que je ne peux pas accepter qu'on parle d'une coquille vide puisque c'est il y a des gens, des gens qui travaillent et qui n'ont jamais cessé de de travailler et je peux vous assurer qu'on qu'on leur donnera tous les moyens nécessaires à évaluer la politique de la ville comme ils l'ont toujours fait et et j'ai d'ailleurs souhaité associer en plus de l'OM TV un un nouveau comité scientifique à la politique de la ville, nommerai un certain nombre des personnes dans les semaines qui viennent, et l'ONPV retrouvera six n'est, si c'est si elle avait réellement perdu toutes ses capacités à faire.

Oui, madame la présidente, monsieur mise chers collègue juste au travers de l'amendement de Madame Artigalas, ce que bien sûr nous allons soutenir il y a la nécessité d'avoir au moment où on veut repartir vers une nouvelle génération de contrat ville l'indispensable nécessité. d'avoir des éléments d'évaluation statistique à la hauteur des cohortes ça été dit aujourd'hui on demande à tous les territoires d'évaluer leurs propres mise en oeuvre des politiques enfin des, des, des contrats de ville qu'ils ont il faut que l'État puisse les additionner les analyser, voir dans quelle direction il fallait que ce soit dans la territorialisation de la nouvelle politique de la ville, que ce soit sur le contenu, les actions, aujourd'hui on ne remet pas en question la qualité des professionnels qui sont à l'intérieur, mais leur nombre, leur quantité les moyens réellement dévolu à avoir une ambitieuse évaluation sans laquelle, comment on peut s'attendre à avoir une politique de la ville, qui évolue dans le bon sens et qui soit adapté aux besoins. Merci, alors je vais mettre aux voix l'amendement 94 qui a reçu, donc un avis défavorable de la Commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient, il est donc adopté alors nous allons procéder au vote des crédits de la mission cohésion des territoires figurant l'je l'je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai 10 minutes, je vous rappelle que la commission des finances s'en remet à la sagesse du Sénat pour le vote des crédits de cette mission. Pardon, monsieur le rapporteur. Abstention personnel c'est ça oui. Je mets aux voix les crédits de la mission. Qui est pour. Qui est pour. Qui s'abstient. Donc ils ne sont pas adoptés. Madame Estrosi Sassone pour l'amendement 373. et je crois pouvoir dire sur l'ensemble des bancs de cet hémicycle et corollairement bien sur la question de la prolongation de la réduction du loyer de solidarité, l'article 41, terre du PLF qui est rattaché à la mission justement pour but de maintenir son rendement à hauteur de 1 virgule 3 milliards d'euros en 2023 l'avenir donc, et donc normalement soumis à la conclusion, on l'a dit, les uns les autres d'un pacte de confiance avec les bailleurs sociaux, sans doute au printemps prochain, est également à la signature de la convention quinquennale avec Action Logement la RLS faut-il le rappeler, a essentiellement été absorbée par les bailleurs sociaux grâce à un accroissement de leur endettement, or aujourd'hui la hausse des taux d'intérêt remet fortement en cause ce modèle ainsi que si la hausse des coûts de production et le parc social est également confronté à un objectif impératif et impérieux de rénovation des logements pour pouvoir continuer demain à les louer, c'est donc la la raison de l'amendement que je vous propose, qui est un amendement qui entend lancer le débat sur la révision de la RLS et enfin connaître ce que le gouvernement entend faire de la RLS à partir de 2023 nous nous pensons tous malheureusement que le gouvernement a l'intention de la prolonger, c'est déjà le cas d'une année supplémentaire, mais que ça pourrait aller beaucoup plus loin et nous pensons que dans cette perspective et surtout dans la perspective de la signature potentiel du pacte de confiance au printemps prochain, il est temps que le gouvernement abattre ses cartes et qui nous disent véritablement ce qu'il entend faire au sujet de la RLS prolongation ou pas, donc on n'a pas l'habitude de demander des rapports, mais cet amendement demande un rapport sous les 4 mois d'ici que le pacte de confiance, soit de Favorable à très favorable à du gouvernement Monsieur le Ministre, c'est ça. Madame la présidente, comme ça a été rappelé, nous sommes dans le le cadre d'un d'un travail partenarial avec le monde HLM et et et le la signature d'un d'un pacte de confiance tous les sujets seront ouverts dans ce travail de pacte de confiance, il y a, il n'y aura aucun, aucun tabou, mais à ce stade, je, je ne vois pas la la nécessité d'avoir ce ce travail d'étude particulier, ça sera donc un avis défavorable. Merci, je mets aux voix l'amendement 73 qui a reçu un avis favorable de la commission défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient donc adopté, je me vois l'article 41 terre qui est pour, contre, que ça tient est adopté après l'article 41 terre 2 amendements identiques, madame la présidente lit tard. Oui, madame la présidente, effectivement, Marie-Noëlle Lienemann, défendra un amendement identique alors le dispositif de l'ARS a pris forme, a pris la forme d'une remise de loyer financés par les bailleurs sociaux pour les locataires éligibles sous condition de ressources à l'APL, en contrepartie d'une baisse concomitante est quasi équivalente comprises entre 90 et 98 % du montant de la RLS des aides personnalisées au logement versées à ces mêmes locataires, si l'on entend la logique d'un tel dispositif à vocation budgétaire puisqu'il permet un virgule 3 milliards d'euros par an d'économies pour l'État sur la période 2000 22022, force est de constater la différence entre la baisse d'APL de 90 à dit à 98 % du montant de l'ARS et la réduction de loyer de solidarité assumée par les bailleurs sociaux fait porter à ces derniers, seule ce coût, le coût de ces 10 à 2 % restants, un rapport de la Cour des comptes du 22 décembre 2020, hé bien recommande de simplifier un tel dispositif peut lisible complexe et qui induit un coût supplémentaire à la charge des organismes de logements sociaux et par ailleurs qui rendent illisible la quittance du locataire, notamment lorsque des opérations de régularisation au type de plusieurs mois passés doivent intervenir, c'est pour ces raisons que le présent amendement propose de fixer la diminution de l'APL versées à hauteur de la RLS perçu, vous comprendrez que derrière cet amendement certes technique et complexe, il y a un vrai enjeu pour les bailleurs et pour les locataires. Merci Madame Lienemann défendu merci l'avis de la commission sur un porteur. C'est une demande d'avis du gouvernement, vous avez l'impression. Merci avait du gouvernement Monsieur le Ministre. Madame la sénatrice je je comprends la la mesure que vous proposez, afin de limiter, si j'ose dire, le nombre d'erreurs relatives au au versement de de la RLS toutefois, si le versement de l'ARS a été source d'anomalies, je crois qu'elles ont été depuis réglés et dans cette optique, je vous propose d'opter pour une stabilisation du système actuel, plutôt que de le faire à nouveau évoluer avec une complexité que vous avez d'ailleurs d'ailleurs vous-même aborder la modification proposée n'il aurait pas la gestion des indus et rappelle au niveau des organismes payeurs puisqu'il y a déjà des régularisations, régulière, sans que l'écart entre la baisse de l'APL et la RLS est un impact particulier le montant de la baisse des APL est déjà très proche légèrement inférieur du montant de la RLS, cet écart de morts cependant nécessaires pour éviter que certains locataires ne soient perdant avec la RLS du fait des tables de calculs ultérieurs ah la formule : je ne rentre pas dans le détail des règles des arrondis, mais pour toutes ces raisons, j'émets un avis défavorable. Merci Madame Lienemann. complexes à décrire, mais complexe, surtout actuellement tels que c'est à mettre en oeuvre pour les organismes, ça leur coûte cher inutilement je soutiens donc cet amendement. Merci, alors je mets aux voix donc l'amendement 1518 pardon, qui a reçu, donc un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour.

Oui merci madame la présidente, alors il s'agit là de différenciation choisir tout simplement dans la mesure où il faut quand même : valoriser le travail de Luchon

joue un rôle essentiel, un rôle de missions d'intérêt général auprès des collectivités d'outre-mer et même auprès des élus parce que quelques fois, ils nous éclairent, ce sont des personnes ressources, le problème de l'habitat social en outre-mer nécessite qu'il y a une réelle volonté de maintenir les actions complémentaires et en synergie avec tous les toutes les instances et tous les acteurs, alors il s'agit de bien vivre ensemble, de travailler tous ensemble parce que là, il se trouve que Lucho ne bénéficient plus des financements qui pourraient lui permettent de jouer son rôle de tirer général alors qu'il est un des signataires du plan logement outre-mer diplôme et porteurs de projets d'intérêt général, il importe que la représentativité de l'action de Luchon soit inscrite au Code de la construction et de l'habitat, pour permettre notamment la continuité des projets de tirer général qu'elle mène avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux qu'elle représente, il faut le savoir, donc il s'agit de dire différenciation et je crois que toutes les actions sont bonnes, donc il ne s'agit pas de faire de différence pour faire

Pour ne pas introduire de de différenciation l'avis du Gouvernement sera défavorable. Merci ma Madame Lienemann, tout aussi efficaces, on nous demande en fait ici d'arbitrer une forme de conflits plus ou moins nette entre une partie des organismes HLM d'outre-mer L Union sociale pour l'habitat, je ne pense pas que ce soit le Sénat qui doivent rentrer dans ce genre de chose je voudrais dire que d'ailleurs tous les organismes HLM ne sont pas adhérents à Luchon et je voudrais quand même noté que le ministre des Outre-Mer invite réellement tous les partenaires, tous les organismes HLM à discuter notamment du nouveau plan logement outre-mer, donc je vous demande de ne pas voter cet amendement. Merci, alors je me vois là et mon 1067, il a reçu donc un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour.

En tout cas, on aura bien compris quelle est la volonté de chacun, alors le supplément de loyer solidarité SLS et appelé de façon anticipée en outre-mer, ce qui crée une inégalité de traitement entre les locataires du parc HLM en outre-mer et en Hexagone, alors il faut savoir que les ultramarins paye cotisent comme tout le monde sauf que dans la réalité, ils ne bénéficient pas des alors que pour le fonds d'aide nationale d'aide à la Pierre et bien tout le monde et tout le monde cotise les activités aussi, par contre, pour en bénéficier, hé bien les ultramarins ne bénéficie pas pour les prêts locatifs aidés d'intégration, donc je voudrais quand même qu'il y ait une réparation de cette injustice et que l'ensemble des cotisants et des Terres territoires qui cotisent puissent bénéficier de cette possibilité d'obtenir des prêts locatifs aidés d'intégration pour les personnes qui le mérite, merci.

Oui, c'est un amendement essentiel qu'on voit la liste des cosignataires et leur qualité, c'est pour aller sur les petites villes de demain avec des crédits dédiés n'ont pas fait chier que la DETR. Je vous remercie beaucoup la vie de la commission, monsieur le rapporteur. qui porte cet amendement s'est beaucoup investi, le rapport à la délégation demande un fonds dédié au programme Petites Villes de demain, et moi j'ai, j'y suis, j'y suis bien sûr favorable alors après il évalue à 2 milliards 7 à regarder en tous les cas, aujourd'hui il y a pas de crédits dédiés à l'investissement dans la petite ville de demain, en revanche, cet amendement ne crée pas le fond cet amendement demande un rapport au gouvernement, et moi je pense que c'est pas par un rapport au gouvernement qu'on va créer le fonds il faut qu'on directement, on fasse une proposition de création d'un fonds dédié aux investissements dans les programmes, petite ville demain, c'est la raison pour laquelle la commission propose un retrait. Si même avis monsieur le Ministre. Même avis retrait ou défavorables. Merci les retirer, merci beaucoup, je vais donner la parole à monsieur le président, Claude Raynal, président de la commission des finances. Oui merci madame la présidente, et merci d'avoir accepté de prolonger un petit peu pour tout le monde vous serait-il possible, que je demande à l'examen séparé de certains amendements de la mission Écologie qui vient cet après-midi pour permettre les regroupements thématiques et éviter une trop longue discussion commune, un sujet qui s'est posé à multiples reprises durant cette semaine voilà. Merci monsieur le président, il y a pas d'opposition, je n'en vois pas, il en est ainsi décidé j'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2023 ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 15 heures 10 pour l'examen de la mission Écologie développement et mobilités durables et la séance est suspendue.